La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 17 décembre 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. J'ai le regret de vous faire part du décès de nos anciens collègues Paul Loridant, qui fut sénateur de l'Essonne de 1986 à 2004, et James Bordas, qui fut sénateur d'Indre-et-Loire de 1992 à 2001.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021. Vendredi dernier, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, dont l'une des missions est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, a activé « le signal rouge » au niveau national. RTE a incité les Français « à réduire leur consommation d'électricité en appliquant des éco-gestes

qu'il se réitère, avec des conséquences peut-être plus graves, d'ici à la fin mars. Pourtant, si le Sénat avait été entendu plus tôt, cet épisode aurait sans doute pu être évité. Depuis bientôt un an, le secteur de l'énergie, et singulièrement le marché de l'électricité, est entré dans une véritable zone de turbulences. Au-delà de son impact sanitaire, la crise de la covid-19 a de graves répercussions sur notre système énergétique. Cette crise affecte lourdement nos énergéticiens, en particulier EDF, car elle réduit le niveau de la demande et des prix des énergies ainsi que la disponibilité des moyens de production. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), « la crise de la covid-19 et les mesures de confinement qui en ont résulté ont un impact hors du commun sur le système énergétique ». Dans ce contexte, dès le 11 juin dernier, RTE a anticipé « une situation de vigilance particulière » pour l'hiver 2020-2021. Cette situation sera d'autant plus critique que les conditions météorologiques seront rigoureuses. Elle s'explique essentiellement par « une disponibilité historiquement basse du parc nucléaire réacteurs de ce parc, neuf seront arrêtés en février et cinq le seront en mars prochain. En effet, la crise de la covid a entraîné des reports dans le programme d'arrêts de tranche d'EDF, c'est-à-dire des opérations de maintenance des centrales. Par ailleurs, certains réacteurs sont indisponibles pour des raisons liées à leur sûreté : Flamanville, Paluel et le Bugey. Pis, d'autres réacteurs ont été arrêtés pour des considérations politiques : avec la fermeture des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, en mars et en juin derniers, le Gouvernement a privé la France d'une puissance de production de 1,8 gigawatt, ce qui représente 1 800 éoliennes de 1 mégawatt ou 15 centrales thermiques de 150 mégawatts. Nous n'avons pas fini d'en payer les conséquences Cette situation de « vigilance particulière » sera très sensible aux mois de février et de mars prochains, de même que dans le Grand Ouest. Je pense en particulier à la région Bretagne, véritable « péninsule électrique » : le déploiement de la centrale nucléaire de Flamanville n'a pas succédé à l'extinction de la centrale à charbon de Cordemais. Cette situation perdurera au moins jusqu'en 2023. Notre parc de production d'électricité est désormais « sans aucune capacité supplémentaire ». En effet, avec les fermetures de centrales nucléaires et thermiques, nos moyens de production se sont réduits, sans être compensés par l'essor des énergies renouvelables (EnR) ou des effacements de consommation. Cette situation se traduira par un recours accru aux centrales thermiques en France, mais aussi à l'étranger. Nous allons dépendre des imports d'énergie de nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, dont- je le rappelle -40 % de la production d'électricité est de source fossile. C'est regrettable pour notre indépendance énergétique, lorsqu'on sait que la France fut traditionnellement exportatrice d'électricité. C'est regrettable pour nos engagements climatiques, lorsqu'on sait que les trois quarts de notre production d'électricité sont entièrement décarbonés. Cette situation ne conduira pas à un complet blackout, c'est-à-dire à une coupure d'électricité à l'échelle nationale, mais elle nécessitera l'activation de mécanismes dits « post-marché », comme l'interruption des consommateurs industriels, la baisse de tension sur le réseau et l'appel aux gestes citoyens.

Les Français sont en droit d'attendre, de la part de leur gouvernement, un diagnostic lucide, des objectifs réalistes et des mesures fortes. Tout d'abord, le Gouvernement doit poser un diagnostic lucide sur la situation que nous traversons. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques, en novembre dernier, Mme la ministre Barbara Pompili avait indiqué que notre vulnérabilité en matière de sécurité d'approvisionnement était liée à la prépondérance de l'énergie nucléaire dans notre mix électrique. Elle avait affirmé que « 75 % de notre électricité est produite à partir du nucléaire », avant d'ajouter : « Quand il y a un raté sur le nucléaire, on en subit les conséquences. C'est la raison pour laquelle il faut diversifier notre mix électrique, afin d'être moins à la merci de ce genre d'aléas en pouvant faire appel à d'autres types de production d'énergie. » Pour ma part, je fais le constat exactement inverse : c'est bien plutôt parce que nous n'avons pas suffisamment investi dans l'énergie nucléaire que nous en sommes arrivés à cette situation. Si les énergies renouvelables doivent être promues- j'en suis le premier convaincu -, elles ne sont pas d'un grand secours pour faire face à la pointe de consommation hivernale, compte tenu de leur intermittence. Faute d'un soutien suffisant à la filière nucléaire, ce sont aujourd'hui des centrales thermiques, de surcroît étrangères, qui tournent à plein régime, non des panneaux solaires ou des éoliennes, soumis aux aléas climatiques. Ensuite, le Gouvernement doit fixer des objectifs réalistes pour sécuriser notre approvisionnement. l'examen du projet de loi Énergie-climat, dont je fus le rapporteur, j'avais regretté le manque d'« anticipation des conséquences de la politique énergétique menée ». Je continue de penser que la fermeture de quatre centrales à charbon, d'ici à 2022, et de quatorze réacteurs nucléaires, d'ici à 2035, aurait dû être davantage évaluée par le Gouvernement, au regard notamment de son impact sur la sécurité d'approvisionnement. En outre, sur l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, le législateur a adopté un objectif d'au moins 6,8 gigawatts de capacité d'effacement d'ici à 2028,

À cet égard, l'interdiction des chaudières à gaz dans les logements neufs, à compter du 1 juillet prochain, issue de la réglementation environnementale 2020, me semble tout à fait prématurée, car insuffisamment évaluée. Enfin, le Gouvernement doit prendre des mesures fortes en faveur de la sécurité d'approvisionnement. La commission des affaires économiques n'a cessé d'avancer des solutions, afin que nous puissions maîtriser la consommation d'énergie l'intensification des appels d'offres en matière d'effacement, le rehaussement du chèque énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique, ou encore le renforcement des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, notamment en matière de régulation et de programmation. Nous avons fait adopter des amendements en ce sens dès le premier collectif budgétaire en mars 2020, mais le Gouvernement n'a conservé aucune de ces solutions de bon sens. Nous avons aussi demandé que le Parlement soit associé aux travaux stratégiques de l'exécutif

est un domaine trop important pour être laissé à des décisions hasardeuses et mal calibrées, car mal évaluées : le risque de blackout que nous subissons nous le rappelle aujourd'hui cruellement. La production d'énergie nucléaire est, en France, un service public, une mission régalienne. En dépendent tout à la fois notre vie sociale, notre vie

2021 : nous souhaitons tous que cette année soit celle de la résilience et de l'apaisement pour tous les Français. Notre pays risque-t-il le blackout électrique ? Notre système de production et d'acheminement d'électricité est-il en mesure de répondre aux pointes de consommation hivernales ? La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim met-elle en danger notre capacité à fournir de l'énergie à toute heure et en tout lieu ?

-que nous risquions un blackout. Je ne crois pas non plus que la fermeture de Fessenheim menace la stabilité de notre système électrique. Au contraire, je crois que l'accroissement des énergies renouvelables contribue à sécuriser notre approvisionnement électrique et que nous utiliserons de moins en moins nos centrales à charbon.

est organisé pour maximiser la disponibilité des réacteurs en hiver. Or la crise sanitaire a contraint EDF à revoir le calendrier de certaines opérations de maintenance. À notre demande, EDF a révisé la planification des arrêts de réacteurs, afin d'améliorer autant que possible la disponibilité du parc en hiver, malgré ces décalages. En outre, nous avons demandé à RTE de mener des analyses prévisionnelles pour évaluer la sécurité de l'approvisionnement électrique au cours des prochains mois.

années, et d'une consommation électrique largement en deçà du niveau habituel à la même époque, en répercussion, malheureusement, des difficultés économiques que traverse notre pays. Je peux donc vous l'assurer : les Français et les Françaises seront approvisionnés sans difficulté. Nous ne risquons aucun blackout. C'est sur le fondement des prévisions de RTE

le volume disponible est doublé grâce aux mesures mises en oeuvre cette année. Ensuite, la consommation de certains industriels peut être momentanément arrêtée : c'est l'interruptibilité, un dispositif auquel les intéressés souscrivent et pour lequel ils sont rémunérés. Si cela ne suffit pas, RTE peut diminuer de 5 % sur de courtes périodes la tension sur les réseaux : les effets d'une telle mesure sont quasiment imperceptibles pour les consommateurs. Enfin- un tel cas de figure reste tout à fait improbable -, en dernier recours, parce que nous sommes aussi préparés aux situations exceptionnelles,

Nous ne serons donc en aucun cas confrontés à des situations de blackout, c'est-à-dire à des coupures massives et non contrôlées sur le réseau. La sécurité de notre approvisionnement électrique est tout à fait garantie.

pour une contribution faible à l'approvisionnement, auraient donc été engagées au détriment du déploiement d'autres capacités de production et de puissance bien plus importantes. Le nucléaire demande de la planification- c'est ce qui a présidé à l'arrêt de cette centrale -, et nous poursuivrons en ce sens. En parallèle, nous utilisons de moins en moins nos centrales à charbon. Les dernières d'entre elles seront arrêtées à l'horizon de 2022, conformément à nos engagements. Nous les employons encore à la marge, comme source d'appoint, pour faire face à des pics de consommation. Pour la période 2019-2020, l'utilisation de ce moyen de production a été sensiblement plus basse que lors de la période 2015-2018. Ainsi, pendant les mois de septembre et d'octobre 2020, cette production a été deux fois plus faible que pendant les années passées. De plus, pendant la période 2012-2018, nous avons fermé 10 gigawatts de capacités de production à base de charbon et de fioul. En aucun cas, la fermeture de Fessenheim ne nous conduit à augmenter notre utilisation du charbon. Notre électricité reste, de fait, la plus décarbonée d'Europe, grâce à notre parc nucléaire, grâce au parc hydraulique et au développement des autres énergies renouvelables. L'épisode actuel nous montre, plus que jamais, la nécessité de diversifier notre mix électrique pour ne pas dépendre d'une seule source d'énergie et pour renforcer la résilience du réseau

les énergies renouvelables contribuent à la sécurité de notre système électrique- les bilans prévisionnels de RTE le confirment -et elles doivent constituer une part croissante de notre mix électrique. L'énergie éolienne a ainsi pu représenter jusqu'au tiers de la production électrique- ce fut le cas le 27 septembre dernier. J'ajoute que cette production est en moyenne plus élevée en hiver, puisque les conditions climatiques s'y prêtent, alors même que la consommation est plus importante.

changement de stratégie ou d'un simple effet de communication, cette décision ne doit pas nous mener à rouvrir des sites de production d'énergies polluantes ou à importer une énergie carbonée de pays voisins en cas de manque sur notre propre réseau. Le nucléaire fait partie des énergies les moins carbonées et reste la plus stable à notre disposition, même si je crois beaucoup aux possibilités qu'offrent les énergies renouvelables, notamment quand elles sont couplées à un stockage par batterie, comme le solaire le prouve. Cette décision ne doit pas non plus fragiliser notre réseau face aux nouvelles consommations électriques.

Fort heureusement, ces besoins nouveaux sont compensés par des innovations permettant de réduire la consommation électrique. Néanmoins, il faut aller plus loin : qu'en sera-t-il en cas de pic de consommation et donc de risques de tensions importantes sur le réseau pouvant entraîner un blackout ? Les véhicules électriques doivent être la solution d'une gestion intelligente du réseau. Ce qu'on appelle le procédé, autrement dit « de la voiture au réseau », est en train d'émerger. La perspective de piloter la recharge des véhicules électriques est source d'espoir et d'efficacité du réseau. Madame la secrétaire d'État, comment envisagez-vous de faciliter l'expérimentation et le développement du pilotage de la recharge des véhicules électriques, dont le potentiel d'innovation pourrait rendre notre réseau plus flexible et prévenir d'éventuels blackouts sur le long terme ? La parole est à

parc nucléaire, qui va bientôt fêter ses quarante ans, représente 77 % du mix électrique français. La voilà, la fragilité de notre modèle, loin des discours rassurants et optimistes : c'est celle d'une énergie coûteuse, fragile, dangereuse et dépassée, qui n'est pas à la hauteur des enjeux de notre siècle le génie français ne serait rien sans son entêtement. Alors que de nombreux pays ont fait le choix de la diversification, nous avons décidé d'investir dans des EPR, comme celui de Flamanville, qui affiche déjà dix ans de retard et dont les coûts sont passés de 3 milliards à 19 milliards d'euros. Quand j'entends que l'on n'a pas encore assez investi dans le nucléaire, j'éprouve quelques doutes La peur du blackout doit permettre à certains d'ouvrir les yeux sur notre mix énergétique : il est urgent de le diversifier pour le rendre plus résilient. Mais la production n'est que la moitié du problème : il faut aussi se pencher sur la consommation et donc sur notre sobriété. Le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire, représente aujourd'hui 45 % de la consommation finale d'énergie en France. La part immense du chauffage électrique, couplée à une grande quantité de passoires thermiques, représente une immense marge de manoeuvre pour faire baisser notre consommation

La loi prévoit une diminution de la consommation d'énergie finale de 20 % à l'horizon de 2030 par rapport à 2012 et une consommation d'électricité stable à cet horizon par rapport à aujourd'hui. En effet, l'électrification croissante des usages doit être compensée par une plus grande efficacité énergétique.

nous disposons des certificats d'économies d'énergie (CEE), du dispositif MaPrimeRénov', qui monte en puissance- vous l'avez vu -, et des aides de l'ANAH, qui constituent le coeur des aides à la rénovation. Les certificats d'économies d'énergie ont été renforcés au printemps 2020 pour la rénovation des logements et locaux tertiaires chauffés au fioul et au gaz notamment, et l'ambition de la cinquième période d'obligation, qui s'ouvrira le 1 janvier 2022, est en cours de définition.

Je constate que le groupe Les Républicains a choisi d'utiliser l'anglicisme « blackout » énergétique. Aussi, je rappelle que, en français, il s'agit d'une coupure généralisée de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie d'un territoire. Cette crainte a été largement relayée par les médias en raison des effets de la crise sanitaire et du confinement du printemps dernier, le calendrier de maintenance du parc nucléaire ayant été retardé avec un nombre anormalement haut de réacteurs à l'arrêt. Le débat de cet après-midi porte donc, d'une part, sur le risque de sous-production par rapport à une demande en forte hausse liée à la chute actuelle des températures et, d'autre part, sur les mesures que prend ou pourrait prendre le Gouvernement pour prévenir un tel phénomène, dans cette période hivernale et de couvre-feu. En France, il est vrai, nous sommes particulièrement consommateurs de chauffage électrique, ce qui peut provoquer une croissance rapide de la demande en énergie au coeur de l'hiver, notamment en début de soirée. Nos voisins connaissent actuellement des froids glaciaux qui pourraient, selon certains scénarios, atteindre notre

Dans ce contexte, pour répondre à une éventuelle surconsommation, des campagnes de sensibilisation sont lancées et des mesures existent en France pour compenser le manque de ressources. de ressources. La plus connue est l'importation d'électricité auprès des pays frontaliers. Toutefois, la situation risque d'être tendue : l'Allemagne est elle aussi concernée par cette vague de froid et sera également soumise à une forte demande sur son réseau intérieur. Dans certains cas extrêmes, RTE peut également demander aux différents gestionnaires du réseau de distribution de réaliser des coupures localisées tournantes de deux heures au maximum. La Bretagne et le sud-est de la France seraient particulièrement touchés par le délestage du fait d'un faible niveau de production d'électricité dans ces zones. Cette possibilité est-elle envisageable ? La parole

d'avoir recours à des délestages, en particulier l'activation des contrats d'interruptibilité des grands consommateurs industriels, permettant à RTE de couper l'approvisionnement avec un très faible préavis,

Il ne s'agit surtout pas de mettre la France dans le noir, mais bien de maîtriser le délestage ciblé d'une partie des consommateurs afin d'éviter des coupures beaucoup plus importantes. Ces opérations font l'objet d'une annonce la veille du délestage. C'est donc sur la base de cet effort volontaire de réduction, des éco-gestes et de ces différentes mesures que nous nous garantissons une absence de blackout. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer en votre nom la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de parlementaires libyens conduite par M. Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants de Libye. La délégation effectue une visite au Sénat à l'invitation du président Gérard Larcher ; elle sera reçue en audience par le président du Sénat aujourd'hui. Le président Aguila Saleh s'exprimera également devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La Libye connaît, depuis 2011, une situation politique, économique et sécuritaire complexe, laquelle affecte au premier chef le peuple libyen, mais aussi l'équilibre de la région et, au-delà, celui du continent européen. Pour y faire face et trouver une issue favorable, la France ne ménage pas ses efforts. La Libye et les Libyens savent qu'ils peuvent compter sur notre appui pour soutenir les efforts de la médiation menée sous l'égide des Nations unies en vue de l'instauration d'un État réunifié, solide, pleinement souverain et de la tenue des élections le 24 décembre 2021. Nous formons le voeu que cette visite conforte les relations entre nos deux pays et contribue à cette sortie de crise en Libye. Nous souhaitons au président de la Chambre des représentants, M. Aguila Saleh, aux parlementaires et à la délégation qui l'accompagnent la bienvenue au Sénat de la République française, ainsi qu'une agréable et fructueuse visite.

Bien que planifiés, la fermeture de Fessenheim en 2020- qui produisait 1 800 mégawatts -et les arrêts de centrales au fioul et au charbon participeront aux tensions de l'offre. En vérité, la centrale de Fessenheim nous manque Si le risque de blackout est maîtrisé cet hiver, il ne peut être écarté à l'avenir, et je remercie les initiateurs de ce débat d'avoir inscrit ce sujet à l'ordre du jour. Il est impératif d'anticiper et d'accroître les marges de manoeuvre, car il n'est pas acceptable de se satisfaire des capacités d'effacement et de coupures d'électricité, aussi courtes soient-elles, comme cela pourrait être le cas au cours du prochain mois. Au-delà de la nécessaire maîtrise de la demande par des gains d'efficacité énergétique, il convient de garantir la stabilité du système électrique. Le développement des capacités de stockage doit s'accélérer, afin d'accompagner les efforts de stabilisation des réseaux. À ce titre, le recours à l'hydrogène constitue un levier de flexibilité pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, ainsi qu'une meilleure intégration des énergies renouvelables. Pour rappel, ces dernières devraient représenter 40 % du mix électrique français en 2030. La stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène, ambitieuse sur le plan financier, avec les 7 milliards d'euros qui lui seront consacrés, évoque timidement le stockage de l'énergie. Plus que celle de la France, les stratégies américaine et britannique accordent une importance particulière à la résilience des réseaux énergétiques au travers du stockage souterrain de l'hydrogène. Dès lors, comment le Gouvernement entend-il accélérer le développement du stockage massif de l'hydrogène afin d'accompagner la transition énergétique et de préserver la sécurité d'approvisionnement de notre pays ?

à court terme, les analyses de RTE n'indiquent pas un besoin de recours à l'hydrogène pour faire face aux pointes de consommation : les sources actuelles de flexibilité sont suffisantes à l'horizon de 2030-2035. Pour autant, l'objectif prioritaire du développement de l'hydrogène est la décarbonation des usages afin de pouvoir l'utiliser directement, notamment dans l'industrie et la mobilité lourde, de manière complémentaire

Nous nous donnons ainsi la possibilité de massifier la production et l'utilisation d'hydrogène, avec une enveloppe de 7 milliards d'euros jusqu'à 2030, dont 2 milliards d'euros consacrons donc des moyens importants au développement de l'hydrogène. Au-delà de 2035, indépendamment du mix électrique choisi, les études montrent un besoin de stockage accru. L'hydrogène pourra alors offrir une solution des plus intéressantes. Plusieurs études prospectives de long terme sont en cours et permettront de quantifier ce besoin et, plus largement, de documenter les enjeux et les leviers de notre futur système électrique, notamment le bilan prévisionnel 2050 de RTE, lequel doit être publié à la mi-2021.

sur les risques de coupure généralisée. En novembre dernier, Mme la ministre Pompili nous confirmait la possibilité de coupures très courtes en cas de grosses vagues de froid. Pour y remédier, il suffirait, selon elle, d'avoir recours à l'effacement, c'est-à-dire de demander aux industries d'arrêter leur production à certains moments, contre rémunération. Or, demain, ce n'est plus seulement aux entreprises électro-intensives que l'on demandera de s'effacer, mais aussi aux particuliers, grâce aux boîtiers Linky. C'est dans cette logique, semble-t-il, qu'EDF a lancé sa scandaleuse campagne #MetsTonPull, alors que 12 millions de personnes sont déjà en situation de précarité énergétique.

Cette injonction à « mettre son pull », discours paternaliste et infantilisant, présupposant que les Français gaspillent, ne saurait en aucun cas masquer votre inertie à développer une politique industrielle ambitieuse pour répondre aux besoins de la Nation. Si la crise épidémique a accentué les menaces sur l'approvisionnement, c'est bien la libéralisation du secteur de l'énergie qui en est à l'origine, et cette situation risque fort de devenir structurelle avec le projet Hercule. Aujourd'hui, des centrales nucléaires et à charbon sont fermées sans que leur apport soit compensé, et les barrages hydroélectriques- les sources d'énergie les plus pilotables et qui permettent d'assurer l'approvisionnement de façon continue, avec le nucléaire -pourraient être confiés, demain, au privé.

en fonction des signaux économiques, c'est indéniable. Dans le cas d'un barrage hydroélectrique à réservoir, ils ont une incitation économique à produire lorsque le prix est plus élevé, c'est-à-dire lorsque s'annoncent des pointes de consommation. Ce système contribue donc à la sécurité d'approvisionnement. Quelle que soit l'option retenue pour le renouvellement des concessions hydroélectriques, ce comportement, dicté par une rationalité économique, ne changera pas. La Commission de régulation de l'énergie, une autorité administrative indépendante, s'assure, par ailleurs, que les acteurs n'abusent pas de leur éventuel pouvoir de marché, et le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, RTE, a la responsabilité d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande sur ce réseau sur ce réseau et peut faire appel aux moyens de production en cas de risque pour la sécurité d'approvisionnement. Un scénario à la Enron, dans lequel un acteur avait pu manipuler le système électrique grâce à la possession de lignes à haute tension cruciales pour la Californie et de nombreux moyens de production, n'est donc pas à craindre en France, et nous y veillerons. Plus largement, ainsi que cela sera évoqué lors du débat dont vous avez demandé l'organisation demain, concernant l'évolution d'EDF, le Gouvernement est très attentif à mettre en place un dispositif dans lequel les concessions hydroélectriques pourront jouer tout leur rôle

À ce jour, un tel déséquilibre ne s'est jamais produit en France. Malheureusement, ce risque ne doit pas être écarté, tant à court terme, avec l'indisponibilité, cet hiver, de centrales nucléaires, qu'à long terme, avec le rééquilibrage progressif du mix énergétique de la France en faveur des énergies renouvelables. Le niveau de ces dernières dans le mix est encore trop faible pour que leur intermittence ait un impact structurel sur le réseau, mais cette problématique devrait se présenter de plus en plus régulièrement à la faveur de leur développement. Quelles solutions peuvent être alors envisagées ? Deux leviers principaux sont à disposition des pouvoirs publics : le dimensionnement des moyens de production pour faire face à des pics de consommation, d'une part, et la flexibilité du système électrique, d'autre part. concerne ce second point, il nous faudra, bien entendu, améliorer les technologies de stockage de l'électricité renouvelable intermittente. En la matière, madame la secrétaire d'État, quelles solutions vous semblent aujourd'hui les plus avancées ? Nous considérons que, à long terme, le développement d'une filière d'hydrogène bas-carbone pourrait contribuer à remédier à l'intermittence saisonnière des énergies renouvelables. L'hydrogène produit en période de surplus d'électricité renouvelable, par exemple en été, pourrait être stocké et retransformé en électricité par le biais de piles à combustible ou de turbines à combustion pendant les périodes de faible production éolienne ou solaire. Le recours au stockage par hydrogène devrait cependant demeurer marginal en France métropolitaine dans les années à venir, en raison du niveau encore modéré des énergies renouvelables

sont suffisantes à l'horizon de 2030-2035. Au-delà de 2035, indépendamment du mix électrique choisi, les études montrent un besoin de flexibilité accru. Plusieurs leviers sont envisageables à cette fin : le développement du stockage, l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'un meilleur pilotage de la demande pour baisser et mieux répartir les pointes de consommation. En ce qui concerne le stockage, l'hydrogène est une option intéressante. Le Gouvernement a mis en place un plan Hydrogène doté de 7 milliards d'euros à l'horizon de 2030 pour massifier la production et l'utilisation de l'hydrogène. À court terme, la priorité du développement de l'hydrogène vise à la décarbonation des usages, notamment dans l'industrie et dans la mobilité lourde. D'autres solutions existent pour le stockage, comme le recours aux batteries au sein du système électrique, de plus en plus fréquent et dont les coûts baissent rapidement. À moyen terme, le développement de parcs de batteries pourra donc apporter cette flexibilité. Le développement des véhicules électriques offre également une opportunité d'améliorer sensiblement la flexibilité du système grâce à des outils de pilotage de recharge. Il est ainsi tout à fait envisageable d'inciter les utilisateurs à charger leur véhicule en milieu de journée, lorsque la production renouvelable est importante, et à restituer en partie cette énergie au réseau le soir, lorsque les besoins sont importants. La parole

De 71 % de production d'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui, ayant, je le rappelle, un impact minime sur le réchauffement climatique et un coût très compétitif, nous devons passer à 50 % en 2035. La marche est très haute et la

à la représentation nationale et à la commission des affaires économiques du Sénat la programmation pluriannuelle des investissements et de leur financement traduisant la planification des investissements et des gros entretiens de production, incluant, bien entendu, les énergies renouvelables La situation actuelle du réseau donne à comprendre que le mécanisme de capacité en place ne répond pas à la couverture des risques identifiés ou constatés. Cette PPI devrait, bien sûr, faire apparaître les investissements planifiés au regard des risques de blackout et des nécessités d'importation en situation de crise de fourniture. Je constate, que le dernier guide public de RTE relatif à la gestion des blackouts remonte à 2004. En quoi le projet Hercule du Gouvernement, en démantelant de fait le groupe EDF, second énergéticien au monde et fleuron de notre souveraineté industrielle, va-t-il améliorer la prévention des blackouts ? Comment va-t-il permettre d'améliorer la résilience de la production et des réseaux de transport et de distribution face aux aléas climatiques et technologiques ? La parole est

ont pu être préparées et nous avons sécurisé notre approvisionnement par un autre mix énergétique, qui nous permet d'aborder sereinement les prochaines échéances, y compris en cas de pic de consommation.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation de « quoi qu'il en coûte » sur le plan économique. Depuis le premier rapport de RTE, au mois d'avril, sur l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité pour l'hiver 2020-2021, nous savons que notre système électrique pourrait être défaillant. Les actualisations de ce rapport font état d'une situation moins alarmante ; pour autant, dans la version du mois de novembre, il est indiqué que la situation fin janvier et durant le mois de février pourrait être difficile si nous subissions une vague de froid. Cela se traduira par le recours à des mécanismes hors marché, qui emportent des conséquences sur l'activité économique. Il s'agit également d'une décision de type « quoi qu'il en coûte » sur le plan des émissions de CO2, car, contrairement à ce que vous nous avez dit précédemment, on ne peut pas vivre uniquement avec des moyens intermittents alors que l'énergie nucléaire est une énergie pilotable et décarbonée.

22 février, avant la crise, et le second en juin. Au début de la crise, le processus de fermeture était, quoi qu'il arrive, déjà engagé de manière irréversible, les travaux nécessaires à la poursuite de l'exploitation n'avaient pas été réalisés EDF ne disposait pas du combustible nécessaire à l'exploitation de la centrale. La situation à laquelle nous avons fait face n'est pas la conséquence de la fermeture de ces deux réacteurs, mais de l'arrêt pour maintenance, d'autres réacteurs de centrales en France. Cela confirme les orientations du Gouvernement sur le besoin de diversifier le mix électrique pour en améliorer la résilience, notamment face à des événements extérieurs tels que nous en connaissons actuellement. Par ailleurs, dois-je vous rappeler le calendrier de l'EPR de Flamanville, dont la mise en service était initialement prévue en 2012 et qui, malheureusement, a pris beaucoup de retard ? Il ne devrait être opérationnel vraisemblablement qu'après la mi-2023.

Certains s'inquiètent aujourd'hui de la survenue d'un blackout énergétique en France. Cependant, un tel scénario ne pourrait se produire qu'en réunissant plusieurs conditions : d'une part, une forte hausse de la consommation d'électricité, elle-même liée à une baisse durable des températures, et, d'autre part, une absence de vent à même d'empêcher le parc éolien de prendre le relais du parc nucléaire.

Des tensions existent déjà au moment des pics de consommation et pourraient bientôt s'amplifier alors que nos capacités de production nationale disponibles lors de ces pointes risquent de diminuer à l'avenir, puisque quatorze réacteurs nucléaires devront être fermés pour atteindre les objectifs fixés par la PPE : une part du nucléaire ramenée à 50 % dans le mix énergétique français d'ici à 2035.

Ajoutons à cette équation le fait que la RE 2020 restreindra de fait l'utilisation du gaz dans les logements neufs, ce qui conduira au retour du chauffage électrique, au risque de solliciter encore plus nos capacités de production d'électricité. d'État, comment pensez-vous concilier, demain, la baisse de la ressource électrique disponible au moment des pics de consommation

progressif et qui ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement. Il s'agit d'un constat appuyé sur des analyses techniques approfondies menées par RTE, intégrant les prévisions d'évolution de la production, de la demande et du fonctionnement du réseau. Pour la production, RTE intègre la modélisation d'un très grand nombre de situations, notamment les aléas météorologiques et ceux qui concernent les moyens de production, comme les retards de maintenance. S'agissant de la RE 2020,

sont évidemment encouragés. Il n'est ainsi pas anticipé d'augmentation de la consommation électrique dans les prochaines années. Concernant les évolutions au-delà de 2035, le ministère de la transition écologique a demandé à l'AIE et à RTE une étude sur les enjeux liés à l'intégration massive d'énergies renouvelables variables dans le système électrique. électrique. Les résultats sont très encourageants et doivent être publiés sous peu. Une analyse plus détaillée de la sécurité d'approvisionnement à l'horizon de 2050 doit être publiée à la mi-2021 par RTE, dans le cadre de son bilan prévisionnel de long terme. Ces études permettront de prendre des décisions

L'orientation qui tend à réduire de façon significative la part des énergies fossiles dans notre production électrique doit être poursuivie et prolongée, en veillant particulièrement à réduire le CO2, principal responsable du réchauffement climatique.

Je souhaite également revenir sur la RE 2020, laquelle prévoit une sortie rapide des énergies fossiles excluant progressivement les chaudières à

du chauffage électrique, notamment des pompes à chaleur

Le ministre Jean-Baptiste Djebbari avait assuré à la représentation nationale que la situation était sous contrôle et qu'il n'y aurait pas de coupure d'approvisionnement. Or, vendredi dernier, RTE a publié un communiqué incitant les Français à à réduire leur consommation pour éviter tout risque de coupure d'électricité. Ce communiqué précise qu'en cas de difficultés d'approvisionnement RTE peut avoir recours à des coupures tournantes.

Madame la secrétaire d'État, au vu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement n'a-t-il pas fermé la centrale de Fessenheim trop tôt, c'est-à-dire avant la mise en route de l'EPR de Flamanville ? En février, la France devrait connaître une vague de froid. Pouvez-vous de nouveau nous assurer que nous serons capables de faire face à cet hiver et aux hivers prochains ? Estimez-vous que votre stratégie énergétique est durable alors que nous émettons beaucoup plus de CO2 en ayant recours au charbon, au fioul et au gaz ?

situation que nous connaissons aujourd'hui résulte d'abord d'une disponibilité moindre du parc nucléaire du fait de différents problèmes de maintenance liés notamment à la crise sanitaire.

Elles sont très simples : les Français vont devoir se rationner. C'est ce que RTE a annoncé jeudi dernier face à la vague de froid qui touche notre pays et à la hausse attendue de la consommation d'électricité. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer ce que nos concitoyens doivent faire lorsqu'ils ont besoin à la fois de se chauffer et de télétravailler ? Comment doit s'effectuer leur choix ? En vérité, cette situation n'est que le résultat de l'imprévoyance du Gouvernement, qui s'apprête à fragiliser notre souveraineté énergétique avec son projet Hercule. Les épisodes de confinement qui ont marqué l'année 2020 et qui menacent de se poursuivre encore en 2021 ont fortement sollicité le secteur énergétique. Si le premier confinement a entraîné une baisse relative de la consommation électrique en raison de la saison et de la baisse d'activité globale, une hausse de 4 % de la consommation électrique des ménages Ces épisodes ont par ailleurs considérablement retardé les opérations de maintenance des centrales nucléaires d'EDF. Je rappelle que, si la France a pour objectif louable de diversifier son mix énergétique, les énergies renouvelables sont encore trop intermittentes pour remplacer le nucléaire, qui assure 70

aux Français le prix de son imprévoyance en exigeant d'eux qu'ils réduisent leur consommation. Risque de surconsommation électrique, d'augmentation du coût des énergies, de conséquences sociales importantes pour les populations déjà durement touchées par le chômage partiel ou la cessation d'activité : quels dispositifs avez-vous prévus pour répondre à tous ces enjeux ?

pour la réplique. J'ai du mal à être convaincu par vos arguments, madame la secrétaire d'État. Si le Gouvernement s'était montré prévoyant, RTE n'aurait pas besoin d'exiger un rationnement de la part des consommateurs. Dans un contexte aussi dur socialement et économiquement que celui que nous traversons, il est injuste de réclamer encore de nouveaux sacrifices aux Français, surtout lorsque ces sacrifices concernent les droits élémentaires à se chauffer et à travailler. À cet égard, le projet Hercule est une épée de Damoclès qui fragilisera et déstructurera notre modèle énergétique, ce qui, au regard des enjeux en termes de souveraineté, n'est pas acceptable.

durant l'hiver en cas de grosse vague de froid. Elle ne possède pourtant pas de boule de cristal ... Elle anticipait simplement son annonce suivante en date du 24 novembre lors de la présentation des principales orientations de la nouvelle réglementation pour la construction des bâtiments neufs, laquelle elle indiquait en filigrane la disparition à moyen terme du chauffage au gaz pour les constructions neuves en fixant un seuil d'émissions de CO2 tellement bas qu'il rendrait presque impossible son installation dans les maisons individuelles à partir de l'été 2021 et pour les logements collectifs à partir de 2024. Ce sont donc désormais presque uniquement des systèmes de chauffage électrique qui seront installés dans tous les futurs logements neufs, accentuant ainsi la tension sur notre système de production d'électricité durant les mois d'hiver. Cela alors qu'il y a presque un an, comme nous le rappelait justement notre collègue Christian Klinger, le Gouvernement fermait la centrale nucléaire encore opérationnelle de Fessenheim, ce qui se traduit désormais par l'émission de 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires en Europe par an. Mais rassurons-nous, mes chers collègues, le 4 décembre, le Président de la République assurait lors de son interview à « Moi, j'assume à fond. Je crois dans l'écologie, je suis pour qu'on soit parmi les champions de la lutte contre le réchauffement climatique. Si on veut réussir, ça veut dire qu'on doit être meilleur encore sur le nucléaire. » Une position réaffirmée le 8 décembre sur le site de Framatome au Creusot.

Plusieurs mesures sont par ailleurs à la disposition du gestionnaire de réseau RTE pour répondre aux pics de consommation que nous pouvons connaître du fait des aléas, notamment climatiques. Le Gouvernement a pris différentes mesures pour accroître leur disponibilité, qu'il s'agisse de l'effacement ou de l'interruptibilité. Pour le long terme, des études sont en cours, entre autres avec l'AIE et RTE, pour fixer les enjeux de notre mix après 2035- les parlementaires y seront bien évidemment associés -, ce qui permettra de définir des stratégies d'investissement dans la production, le réseau, le stockage sans oublier la maîtrise de la demande, en tenant compte des enjeux de sécurité d'approvisionnement. Concernant la RE 2020, un travail fouillé est conduit pour affiner les détails des obligations- leur niveau et leur date d'entrée en vigueur. L'amélioration de la performance des bâtiments permettra de déployer

Depuis septembre aussi, du fait de l'arrêt de cette centrale nucléaire, il arrive à EDF de devoir importer très cher de l'électricité produite au gaz ou au lignite en Allemagne. Ainsi, hier, pendant vingt-quatre heures, la France a importé l'équivalent de six tranches nucléaires. Ces mesures successives et l'intermittence hivernale de l'éolien et du solaire, presque absents de la production électrique française, mettent en danger notre réseau. S'ajoutant à l'incapacité d'EDF de tenir les délais de livraison du futur réacteur de Flamanville, ces difficultés fragilisent la sécurité de l'approvisionnement électrique. Jeudi dernier, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, RTE, a demandé aux Français de réduire leur consommation d'électricité face à un risque de tension sur notre réseau. Le risque de coupure chez les particuliers n'est pas un acte banal : la France ne saurait s'y habituer. Face au risque d'instabilité de notre réseau électrique dû à notre dépendance envers les autres pays européens et à nos orientations énergétiques, quel est le nouveau calendrier pour la mise en service du futur réacteur de l'EPR de Flamanville ? La parole est ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Sido, le Gouvernement porte une attention particulière au calendrier de mise en service de ce réacteur. Les essais à chaud se sont terminés en février 2020. Les premiers assemblages de combustible ont été approvisionnés en octobre pour être entreposés, le processus de remise à niveau des soudures situées sur le circuit secondaire se poursuit, le scénario de reprise des soudures de traversées de l'enceinte étant en cours d'examen par l'ASN (Autorité de sûreté nucléaire). Malgré la crise sanitaire, EDF n'a pas fait

4 novembre 2006, 15 millions de foyers ont été privés d'électricité, dont 5,6 millions en France, du fait d'un incident en Allemagne.

Nous partageons tous l'objectif de consommer moins d'énergie et de la consommer mieux, en particulier quand elle est d'origine fossile. Si la demande faite aux Français de réduire leur consommation était sans doute nécessaire compte tenu des ressources disponibles, elle résonne avant tout comme un aveu d'échec, ou en tout cas d'impuissance à réguler les flux de notre mix énergétique au sujet duquel les orateurs précédents sont intervenus. Au moment où nous nous orientons fortement et positivement vers une économie décarbonée reposant sur le tout-électrique- dans les transports, dans le bâtiment aux besoins croissants du numérique, comme nous le verrons dans quelques minutes lors de l'examen de la proposition de loi de Patrick Chaize -, il me paraît nécessaire d'aborder sans dogmatisme la question de l'origine de l'énergie indispensable au fonctionnement de notre pays dans tous ses usages. Les Françaises et les Français n'ont pas à subir les atermoiements successifs des décideurs publics et les conséquences des décisions arbitraires- parfois démagogiques -qui nous ont conduits à cette situation potentielle. Cela ne serait pas digne d'un grand pays comme le nôtre. Du bon sens, du réalisme, du pragmatisme, une vision : tel est mon voeu à l'aube de cette nouvelle année, madame la secrétaire

La politique énergétique du Gouvernement permettra un système électrique plus diversifié. C'est une des clés de la résilience face aux aléas que nous ne connaissons malheureusement que trop aujourd'hui. Les tensions sur la sécurité d'approvisionnement de cet hiver illustrent le risque d'un système qui reposerait massivement sur une seule technologie.

nous sommes attachés. Ce constat s'appuie sur des analyses techniques approfondies, menées notamment par RTE, qui intègrent les prévisions d'évolution de la production, de la demande et du fonctionnement du réseau. Pour la production, RTE intègre la modélisation d'un grand nombre de ces situations. Au-delà de

de sécurisation de ce mix énergétique et de notre sécurité d'approvisionnement. Concernant la question essentielle de la décarbonation, RTE a estimé que le parc solaire et éolien a permis d'éviter en 2019 l'émission de 22 millions de tonnes de CO2 au niveau européen, soit les émissions annuelles d'environ 12 millions de véhicules.

La loi de 2015 relative à la transition énergétique a marqué un tournant dans la politique énergétique française en prévoyant la réduction à l'horizon de 2025 de la part du nucléaire dans la production d'électricité à hauteur de 50 %, objectif reporté à 2035 depuis la loi Énergie-climat car totalement irréaliste. Voilà comment, par dogmatisme, on réduit notre capacité de production électrique pilotable et propre, à savoir le nucléaire, pour la remplacer par des énergies tout aussi propres mais intermittentes et aléatoires, à savoir les énergies renouvelables, avec comme conséquence l'incapacité de couvrir la consommation des ménages et des entreprises en électricité en cas d'hiver rigoureux, et ce peut-être dès cet hiver. Le Gouvernement veut s'appuyer sur l'électricité d'origine renouvelable pour pallier la réduction de la production d'électricité d'origine nucléaire, mais les voyants sont au rouge les objectifs de la politique énergétique nationale risquent de ne pas être atteints et le compte d'affectation spéciale « Transition énergétique », qui assurait le financement des EnR, a été supprimé du budget. Les dispositifs de soutien aux EnR sont entrés dans une zone de turbulences, puisque la baisse des prix des énergies renchérit les charges de service public de l'énergie qui les sous-tendent. L'hydroélectricité, première source d'énergie renouvelable en France, est menacée par la demande d'ouverture à la concurrence du secteur par Bruxelles. En tout cas, les projets sont à l'arrêt. Les EnR sont aussi le parent pauvre du plan de relance. Au total, 28 % des objectifs fixés par la PPE d'ici à 2023 ne sont pas réalisés pour les installations photovoltaïques, éoliennes et hydrauliques. secrétaire d'État, quelle est donc la stratégie pour le développement des EnR électriques ? Seront-elles un jour suffisantes pour pallier le recul de l'électricité nucléaire dans le mix énergétique et assurer la continuité du service ? Bravo

Pour atteindre cet objectif, nous déployons des dispositifs de soutien public en faveur des énergies renouvelables. En 2021, plus de 6 milliards d'euros seront consacrés à ce soutien. Grâce à cet effort soutenu depuis plusieurs années, la compétitivité des énergies renouvelables, notamment électriques, s'est fortement améliorée.

nous travaillons effectivement sur tous les leviers : nous avons mis en place un calendrier des appels d'offres pluriannuel, qui donne aux acteurs une visibilité leur permettant de développer leurs projets et leur stratégie ; nous soutenons l'innovation par le PIA pour développer les technologies et des appels d'offres spécifiques pour les déployer ; et nous travaillons sur des questions de planification et de délais de raccordement, de qualité de la concertation des projets et de planification jusque dans l'appropriation locale, qui constitue un enjeu fort dansnos territoires. Les études techniques approfondies qui sont menées par RTE montrent que la diversification du mix électrique électrique prévue par la loi, en particulier dans le cadre du programme de fermetures de réacteurs et du développement des énergies renouvelables, ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement à moyen terme. Ces évolutions seront évoquées dans l'étude qui doit être publiée mi-2021 par RTE, notamment sur cette sécurité d'approvisionnement. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comment en est-on arrivé là ? C'est sans doute la question qui est venue à l'esprit d'un certain nombre d'entre nous lorsque RTE a demandé aux Français, vendredi dernier, de réduire leur consommation pour éviter des coupures d'électricité sur le territoire.

dernier, la situation climatique était-elle si rigoureuse et les besoins prévisionnels étaient-ils si exceptionnels que nous devions craindre à ce point un blackout ? En réalité, non ! Les températures affichaient seulement quelques valeurs légèrement négatives et le pic de la demande était estimé à 88 gigawatts, très loin du maximum historique du 8 février 2012 à hauteur de 102 gigawatts.

le pétrole dont notre sol national est quasiment dépourvu, mais d'une énergie pour laquelle notre pays a savamment construit une stratégie d'autonomie dès les années 1960. Hélas, l'absence de décisions anticipatrices et les renoncements sur l'autel des petits arrangements politiques ont mis à mal cette souveraineté, basée sur une avance technologique reconnue dans le domaine du nucléaire Certains, dont la ministre de la transition écologique, évoquent la possibilité de se tourner radicalement vers d'autres sources d'électricité et caressent même l'espoir d'un mix totalement renouvelable à l'horizon de 2050. 2050. D'autres sont nettement plus sceptiques et partagent l'analyse de l'ancien député socialiste Jean-Yves Le Déaut, qui déclarait en 2017, en sa qualité de président de l'Opecst Le développement de la puissance éolienne et photovoltaïque installée ne contribue pas à assurer la sécurité d'approvisionnement, en tout cas pas dans la période de pointe la plus critique, celle du soir.

Quels que soient les rêves des uns et des autres, la géographie naturelle de la France n'est pas celle de la Norvège. Elle ne permet pas de remplacer notre capacité de production par des sources intermittentes et non pilotables. Au contraire, et il faut avoir le courage de le dire aux Français, nous importons régulièrement de l'énergie très fortement carbonée, en raison notamment de la baisse de notre production d'origine nucléaire, liée à la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim. Certes, plusieurs pistes prometteuses ont été mentionnées au cours de ce débat, des systèmes de stockage par batteries à la production d'hydrogène vert, mais dans le même temps on abandonne le programme Astrid sur les réacteurs nucléaires de quatrième génération, alors que d'autres pays accélèrent

Ces mesures se traduisent par le développement de solutions consommatrices d'électricité, au premier rang desquelles les pompes à chaleur. Par ailleurs, une récente étude du cabinet E-CUBE et de l'Institut d'économie de Cologne montre qu'une vague de froid rigoureux en Europe pourrait conduire à un déficit de capacité de production

Déjà fragilisée par la fin brutale de la saison 2019-2020, du fait du premier confinement et d'un été en demi-teinte, la filière de la montagne va subir de nouvelles pertes économiques sèches, ce que reconnaît d'ailleurs le juge des référés du Conseil d'État dans son ordonnance du 11 décembre 2020.

Il est maintenant temps d'écouter la demande formulée dès le début par les acteurs de la montagne : qu'une date de reprise d'activité soit fermement fixée et que l'on s'y tienne, ou bien que l'on nous dise si nous allons vers une saison blanche. Il n'est plus possible de continuer à tenir l'ensemble des acteurs économiques de la montagne dans l'obscurité.

Opérateurs de remontées mécaniques, commerçants, professionnels de l'immobilier, collectivités territoriales ou travailleurs indépendants comme les médecins ou les pharmaciens, tous sont concernés. Sans la fréquentation touristique française et étrangère, l'économie de montagne est à l'arrêt. Les taux d'occupation des stations atteignent à peine les 10 % pour les plus touchées, et les domaines skiables ont déjà perdu entre 20 % et 30 % de leur chiffre d'affaires annuel durant la seule période des vacances de fin d'année. La décision du Gouvernement va donc compromettre durablement les capacités d'investissement de l'ensemble des acteurs de la montagne. La filière d'excellence des sports d'hiver anticipe une baisse des investissements de 50 %. En outre, les aides mises en place par le Gouvernement ne suffiront pas à pallier les difficultés liées à la fermeture

existants pour limiter la propagation du virus et les accidents, mais ne laissez pas à l'abandon cette économie, qui, en raison de ses spécificités, ne pourra pas reprendre une activité normale au printemps ministre les principales propositions que nous avions formulées. Il est resté sans réponse à ce jour ; je le tiens à votre disposition. Au nom de l'ensemble des acteurs de la montagne, je vous prie de faire le bon choix et de permettre une reprise d'activité le plus rapidement possible. Deux mesures me paraissent particulièrement intéressantes à mettre en oeuvre, sans débourser 1 euro : d'une part, étaler les vacances d'hiver sur six semaines au lieu de quatre, afin de soutenir l'activité des stations sur les « ailes de saison d'autre part, envisager de différencier les restrictions selon les départements, comme c'est le cas actuellement pour le couvre-feu, en observant le taux moyen d'occupation des lits d'hôpitaux. Les stations des départements situés au-dessous d'un certain seuil pourraient alors être autorisées à rouvrir leurs remontées mécaniques. J'espère que vous envisagerez sérieusement ces propositions. La possibilité de cette différenciation me conduit au second point de mon propos : il faut continuer d'avancer sur le chemin d'une meilleure adaptation des normes législatives et réglementaires aux spécificités des territoires de montagne et des massifs. Ce travail doit commencer dès la conception de ces normes.

renforcer les liens avec le Conseil national d'évaluation des normes et le Conseil national de la montagne, ou bien encore à prévoir des expérimentations spécifiques. Pour répondre à la Pour répondre à la désertification médicale, il me semble nécessaire de modifier le fonctionnement et la gouvernance des agences régionales de santé, de favoriser le développement de l'offre de stages en ambulatoire dans les zones de montagne, de développer la création de maisons de santé pluriprofessionnelles et de garantir le maintien d'une offre hospitalière de qualité, en proximité. L'accès territorial au numérique et la lutte contre l'illectronisme sont d'autres sujets prioritaires. Le Gouvernement s'est fixé des objectifs ambitieux, qu'il est plus que jamais nécessaire d'atteindre. Enfin, des questions d'attribution de compétences se posent, en particulier pour l'eau et l'assainissement. Une proposition de loi a été récemment déposée à ce sujet. L'adaptation des territoires de montagne au réchauffement climatique remet durablement en cause leur modèle économique. Cette problématique a été peu abordée par les précédentes lois Montagne, alors qu'elle est vitale pour nos territoires, surtout pour les stations de basse et moyenne altitudes. Pour rappel, depuis les années cinquante, les températures annuelles moyennes dans les Alpes ont augmenté de deux degrés. Si le risque de disparition des sports d'hiver est limité à l'horizon de 2040-2050 pour les stations situées au-dessus de 1 800 mètres d'altitude, elles seront confrontées comme les autres au manque d'enneigement, en particulier sur les « ailes » de la saison hivernale. Cette situation est très préoccupante, car la viabilité d'un domaine skiable suppose une durée minimale d'ouverture de cent jours par an. Certes, des outils existent pour sécuriser l'enneigement, comme la neige de culture. Nous devons cependant trouver des solutions pérennes, écologiques et moins coûteuses pour les stations, notamment les plus petites.

d'abord, il faut accompagner les territoires de montagne dans le développement d'un tourisme « 4 saisons » ou « 2 saisons plus », ainsi que dans la diversification des activités touristiques, qu'il s'agisse du VTT, de la randonnée, de l'escalade, du parapente, des loisirs en eau vive,

Le concours de l'État et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui dispose depuis peu d'un programme spécifique pour la montagne, sera déterminant pour aider les collectivités à construire et à faire aboutir leurs projets. Ensuite, cette transition doit être soutenue et accompagnée sur le plan financier. Il est donc nécessaire de créer un fonds spécifique d'adaptation au changement climatique en zone de montagne, pour restructurer les activités économiques face au recul de l'enneigement et financer la réhabilitation énergétique de bâtiments touristiques.

la politique de la montagne vise l'équilibre entre la préservation d'un patrimoine naturel exceptionnel et le développement économique. Elle doit aussi adapter la gouvernance de ces territoires à leurs spécificités.

Je côtoie les élus de montagne depuis le début de mon engagement dans la vie publique. Nous avons noué entre nous une forme de solidarité transpartisane qui fait notre force. Les élus de la montagne sont inventifs et ingénieux, de sorte qu'ils trouvent souvent avant les autres des solutions à des problèmes qui se posent sur le reste du territoire.

soumis à des contraintes naturelles plus fortes qu'ailleurs, les élus de la montagne redoublent de ténacité et de persévérance. Ils savent mieux que quiconque ce que veut dire le proverbe « Aide-toi, le ciel t'aidera », qui est toujours préférable à « Tout ce qui tombe du ciel est béni », car le ciel est souvent un peu trop parisien Vous comprendrez donc aisément que, dans mes fonctions actuelles de secrétaire d'État chargé de la ruralité, j'aie un fort tropisme pour la montagne. Certains esprits malicieux m'avaient d'ailleurs qualifié, dès ma nomination, de « secrétaire d'État à la montagne Je ne récuse nullement cette qualité, même si j'ai vocation à traiter tous les sujets de la ruralité et pas seulement ceux où il y a « de la pente » ! Je suis aussi chargé de suivre la mise en oeuvre de l'agenda rural, ce grand plan national en faveur de la ruralité, dont les 181 mesures profitent directement aux territoires de montagne. Cependant, ce débat couvre un champ plus large, car la montagne n'est pas que rurale. Les territoires de montagne se caractérisent par leur grande diversité. Parmi les sujets que nous allons évoquer, beaucoup débordent le périmètre du ministère de la cohésion des territoires auquel mon secrétariat d'État est rattaché. Il s'agit notamment des sujets agricoles ou encore des aides compensatrices des conséquences de la crise de la covid. Je m'efforcerai néanmoins de répondre à toutes les questions, et pour celles qui ne relèvent pas du ministère de la cohésion des territoires ou pour lesquelles je n'aurais pas tous les éléments à ma disposition, je m'engage à vous apporter le cas échéant des compléments par écrit, à l'issue du débat.

Tous nos espoirs reposent désormais sur l'efficacité du vaccin. De longues semaines de privations sont, hélas, encore à venir. Je sais mieux que quiconque ce que cela implique pour les stations de montagne.

Ils réalisent habituellement un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,4 milliard d'euros par an, dont l'essentiel dans un intervalle de quatre à cinq mois en période hivernale, alors que les coûts qu'ils supportent sont répartis sur l'ensemble de l'année.

Je précise qu'il sera évolutif au cas où de nouvelles périodes de confinement s'avéreraient malheureusement indispensables. Il faut préserver l'avenir en la matière. L'ensemble des commerces situés dans les stations de ski et les vallées qui en dépendent

La mesure s'applique non seulement dans les communes des stations de ski, mais aussi dans celles des vallées qui en dépendent : communes de montagne, membres de l'EPCI support d'une station de ski et n'appartenant pas une unité urbaine de plus de 50 000 habitants.

Les moniteurs de ski, à titre individuel, peuvent accéder au fonds de solidarité, avec un droit d'option leur permettant une compensation des pertes de recettes allant jusqu'à 10 000 euros ou 20 % du chiffre d'affaires réalisé sur la même période en 2019. Les autres activités touristiques et les activités hôtelières liées au fonctionnement des stations de sports d'hiver bénéficient déjà d'une aide renforcée du fonds de solidarité, grâce à leur intégration au plan Tourisme. Enfin, afin de permettre aux professionnels de la montagne de sécuriser les embauches des saisonniers, le Gouvernement a décidé, dès le 30 novembre dernier, d'octroyer le bénéfice de l'activité partielle aux entreprises concernées, jusqu'à la reprise d'activité dans les stations.

Nous sommes, hélas, contraints à la plus grande prudence, à l'heure où de nombreux pays reconfinent et où l'on ignore encore l'état précis de diffusion de nouveaux variants sur le territoire national. Les propositions que vous formulez doivent être étudiées. Le Gouvernement doit rester à votre écoute. Il le fera, et je continuerai d'être votre interlocuteur. Cette crise agit aussi comme un révélateur. Elle met en lumière la forte dépendance de certains territoires à un type d'activité. Nous devons donner aux collectivités qui le souhaitent les moyens d'y remédier et de s'adapter. C'est tout le sens du programme Montagne que nous concevons avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. Il s'agit du premier programme national depuis le plan Neige des années 1960-1970. Une consultation des acteurs de la montagne est en cours à ce sujet et se déroule dans le cadre du Conseil national de la montagne, d'une part, et des comités de massif, d'autre part. Ce programme privilégiera le « cousu main ». Il ne reposera pas sur des appels nationaux à manifestation d'intérêt conçus depuis Paris. L'idée est de construire des projets qui partent des territoires et d'apporter l'aide nécessaire, notamment en matière d'ingénierie. La contribution du Sénat, au travers de ses travaux et des échanges que nous avons, sera évidemment déterminante. Je n'oublie pas non plus que, dans son rapport public annuel de 2018, la Cour des comptes a appelé les collectivités à faire évoluer rapidement la gouvernance et le fonctionnement des domaines skiables, pour s'adapter suffisamment tôt à un avenir où le ski et les sports de neige ne seront plus leur seule ressource.

interactif, la parole est à M. Guillaume Gontard. À l'heure où l'absence de perspectives met les professionnels et les communes de montagne à l'agonie, à l'heure où la région des Alpes du Nord est celle qui se réchauffe le plus en France, à l'heure où notre plus grand réservoir naturel d'eau s'assèche, notre responsabilité à l'égard des territoires de montagne est immense. La crise à la fois économique et écologique que nous traversons a sonné le glas d'un modèle qui voudrait à tout prix maîtriser le développement de la montagne en gommant ses aléas, ses aspérités et ses aménités. En réalité, cette situation d'exception pourrait offrir l'opportunité de montrer tous les atouts de nos territoires de montagne, dont les capacités de résilience sont considérables. En effet, au-delà d'une aire de jeux, les massifs montagneux les massifs montagneux constituent d'abord un réservoir de biodiversité extraordinaire et une ressource hydrologique majeure. Or les scientifiques sont formels : d'ici à la fin du siècle, la plupart des glaciers situés au-dessous de 3 500 mètres d'altitude auront disparu. Agissons pendant qu'il en est encore temps, avant que ces territoires ne deviennent suraménagés ou sanctuarisés ! Parmi les Français, 90 % considèrent que la montagne est un atout pour le pays. La fréquentation inédite des sites de montagne après les périodes de confinement montre leur attachement à la nature et leur besoin de grands espaces. De nombreux touristes ont découvert, cet hiver, la montagne autrement. Appuyons-nous sur les femmes et les hommes qui participent au quotidien à la vitalité des territoires de montagne, maintiennent les liens de solidarité, construisent un modèle économique plus durable, plus juste et plus respectueux de son environnement Il est urgent que nous nous dotions d'une politique de la montagne à la hauteur des enjeux écologiques, sociaux et économiques. Nous ne pouvons pas réduire l'avenir des territoires de montagne à la seule question de la diversification touristique, comme le propose l'ANCT. Monsieur le secrétaire d'État, il est urgent de bâtir une véritable politique de transition des territoires de montagne avec les moyens consacrés. La

et plus respectueux de l'environnement particulièrement fragile des zones de montagne. Nous allons travailler sur l'idée commune d'un fonds de résilience du tourisme en montagne, qui pourrait s'adosser au programme Montagne, de façon à associer relance et transition écologique.

inspirante. La parole est à M. Bernard Buis. En tant que parlementaire de la Drôme, où les Préalpes constituées par les massifs du Royans et du Vercors s'élèvent sur les contreforts, je me réjouis de ce débat sur la montagne. la problématique que je soulève concerne le droit de l'urbanisme dans ces communes. Je sais que nombre de maires, souvent de petites communes, attendent votre positionnement et votre vision sur ces territoires. Aujourd'hui, les documents à l'initiative des municipalités sont la carte communale ou le plan local d'urbanisme. Si ce cadre convient sans doute aux villes et aux communes de plus grande taille, vous savez aussi que ce sont des documents longs à élaborer et avec de forts risques de contentieux, notamment pour les PLU. De plus, la procédure inclut la concertation et la consultation des services associés, ainsi que la vision de l'État, notamment pour ce qui concerne la constructibilité dans des secteurs agricole, forestier ou naturel. Considérant ces procédures non seulement coûteuses, fastidieuses, mais aussi fragiles juridiquement, le résultat est aussi contraignant pour adopter une vision communale de la constructibilité. C'est pourquoi de nombreuses communes de montagne sont régies par le règlement national d'urbanisme en l'absence d'autres documents arrêtés par la municipalité, et les autorisations d'urbanisme sont signées par les maires au nom de l'État. Là, nous constatons des disparités d'appréciation. En effet, les services instructeurs se rendent rarement sur site pour apprécier la continuité de construction, et le maire peut être en désaccord sur l'avis rendu. J'ai encore en mémoire le refus de permis de construire distillé par la DDT de la Drôme à la commune de Montclar-sur-Gervanne sur un quartier, pour pour un pétitionnaire, alors que trois maisons avaient auparavant été construites avec autorisation, la commune ayant déjà assumé la mise en place des réseaux secs et humides, avec logettes et regards installés en bordure des propriétés.

montagne »- je reprends là ce qu'a dit Cyril Pellevat -dans la loi 4D. Pour les petites communes, le règlement national d'urbanisme offre des possibilités d'aménager le territoire pour des besoins ponctuels. La continuité de l'urbanisation constitue évidemment un critère essentiel, apprécié, au cas par cas, par les services de l'État.

moi, monsieur le secrétaire d'État, il y a des économies touristiques meurtries après ces vacances de Noël, mais surtout des vies quotidiennes locales qui sont bouleversées, sans perspectives réalistes d'ouverture avant quelques mois.

Je demande une indemnisation prolongée et une réflexion de moyen terme sur le statut des saisonniers et loueurs, qui pourraient bénéficier de formes coopératives ou de portage salarial. À côté de ces mesures immédiates, il est sans nul doute indispensable d'accélérer la mutation des stations, afin d'anticiper concrètement les effets du réchauffement climatique sur nos massifs et nos vallées. La montagne doit pouvoir s'apprécier en toutes saisons, ce qui va nécessiter des investissements de long terme. Or nos communes et collectivités, extrêmement dépendantes des ressources touristiques ou du thermalisme, alors qu'elles sont essentielles pour absorber l'onde de choc de 2021 et transformer durablement notre modèle économique et social,

et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale ». Comment allez-vous soutenir un effort supplémentaire au bénéfice de collectivités locales aujourd'hui dépourvues de ressources pour entretenir la montagne, notre bien commun, et faire vivre dignement ses habitants au cours de ce premier semestre de 2021 ?

la montagne, vous l'aimez, et, en ce sens, il est heureux que vous représentiez le Gouvernement cet après-midi. Je veux profiter de ce débat initié par le groupe Les Républicains pour vous alerter sur la situation financière des communes et intercommunalités de montagne à l'horizon de 2021 et 2022. Bien sûr, je ne méconnais aucun des efforts consentis par l'État pour maintenir un niveau de ressources aux collectivités territoriales en général. Le Sénat a d'ailleurs pris toute sa part à cet effort. Les communes touristiques de montagne sont en train de vivre un double traumatisme. il y a cet hiver, avec une activité drastiquement réduite et la perspective de voir leur budget fondre comme neige- elle est pourtant abondante cette année -au soleil. Mais, sur un tableur de Bercy, ces communes apparaissent comme ayant un niveau élevé de dépenses, en fonctionnement comme en investissement, pour un nombre d'habitants permanents relativement faible. faible. La spécificité de certaines recettes fiscales ou non fiscales rend la situation encore plus difficile à appréhender. Autrement dit, ces communes aux finances dynamiques sont considérées comme riches.

auront besoin d'un suivi individuel et d'un accompagnement spécifique, avec des mesures, qui ne peuvent pas être les mesures prévues dans les différents PLFR ou dans le PLF pour 2021. pour 2021. Êtes-vous en mesure d'apporter des réponses de nature à rassurer ces collectivités et les EPCI auxquelles elles appartiennent ? La parole est

raquette. Plus de 300 communes de montagne ont donc reçu un acompte en novembre. Le calcul définitif et individualisé pour 2020 aura lieu avant le 31 mai. Je m'arrête là, sinon je vais dépasser mes deux minutes

Cette activité saisonnière est indispensable au bon fonctionnement des entreprises du tourisme, notamment les stations de ski. Un travail de fond doit être mené pour accompagner ces territoires vers un « tourisme 4 saisons », dans une stratégie globale d'adaptation au changement climatique et de fidélisation des compétences saisonnières. Le Conseil d'État a sanctionné deux dispositions très contestées de la réforme de l'assurance chômage et mis en avant le caractère profondément injuste de cette réforme. La plus controversée de ces dispositions, pour les demandeurs d'emploi, est le changement du mode de calcul de l'allocation chômage. Les nouvelles règles de ce régime impacteront fortement les saisonniers et la pérennité économique de nombreux systèmes d'activité de montagne. En effet, c'est en montagne que les activités sont les plus dépendantes des saisons. Notre groupe demande, depuis son instauration, le retrait de cette réforme. Avec la crise de la covid-19, c'est plus de 1 million de saisonniers qui ont perdu leur source de revenus et seront, de surcroît, victimes des effets de cette réforme du chômage. Les Les pistes envisagées jusqu'à maintenant sont foncièrement insatisfaisantes, alors même que de nombreux Français en difficulté sont déjà très durement touchés par les conséquences de cette crise. De plus, nous ne sommes pas à l'abri que cette situation sanitaire perdure, voire réapparaisse dans un avenir plus ou moins proche. Les solutions qui s'imposent sont l'adoption d'une année blanche pour les saisonniers, extras déterminée d'usage, et l'abandon de la réforme du chômage. À quand ces annonces, tant espérées dans nos massifs ? À quand une réelle réflexion sur le statut de saisonnier ?

et de construction pour les communes situées en zone de montagne. Si les deux lois Montagne ont permis d'élaborer des mesures spécifiques à ces communes, afin de leur permettre une différenciation avec les zones rurales du reste du territoire, il existe actuellement des problèmes en matière de constructibilité, qui nuisent au bénéfice initial établi par le législateur. Le rapport d'évaluation de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur les lois Montagne évoque même une « asphyxie des possibilités de construction en montagne ». Certaines communes ne se voient ainsi délivrer qu'un unique permis de construire par mandat municipal, face à une administration toujours plus tatillonne, alors que des aménagements nécessaires à la vie quotidienne et au développement économique sont attendus. Je voudrais aussi vous saisir,

par exemple, que la nouvelle construction soit un peu différente de celle qui a été détruite, à travers une surélévation ou encore un déplacement sur la même parcelle

La situation est grave. Nous avons besoin de concertation entre les niveaux local et national, de visibilité sur l'ouverture des remontées mécaniques et de solutions dans un futur très proche. Les territoires de montagne sont sous tension, alors qu'ils sont déjà soumis à des problèmes chroniques d'ampleur. Nous faisons face à une désertification multiple, notamment médicale. L'accès aux soins ne doit pas être un luxe, surtout dans la situation actuelle. Nous avons des problématiques liées aux réseaux, qu'ils soient de transports ou de télécommunications. Nous vivons une autre désertification, moins médiatique, certes, mais aux conséquences importantes sur l'écosystème des territoires de montagne : en matière d'agropastoralisme, nos jeunes ont du mal à s'installer et nos agriculteurs actuels peinent à résister. Nous observons une véritable perte de vocation de berger. C'est un savoir-faire, une filière et des traditions qui risquent de disparaître. Nous allons vers une crise économique, humaine et écologique. Au cours des vingt dernières années, nous avons perdu 50 % de nos surfaces d'estives et de pâturages. Leur remplacement par des taillis ne fera qu'accroître les risques d'incendie. les risques d'incendie. Le pastoralisme est un équilibre fragile entre l'homme, l'animal et le milieu ambiant. Quelles mesures incitatives comptez-vous mettre en oeuvre, afin de préserver les bienfaits économiques, écologiques et sociaux de ces activités dans nos montagnes ?

Cette fermeture, compensée par de très maigres dérogations, pénalise tous les acteurs de la montagne. Dans mon département des Hautes-Alpes, que Joël Giraud connaît bien, l'annonce de la fermeture administrative des remontées mécaniques s'est traduite par une diminution des réservations de près de 71 % par rapport à l'année dernière. Cette situation devient intenable pour les domaines skiables bien sûr, mais aussi pour les commerçants, les hébergeurs, les saisonniers, les entrepreneurs de l'événementiel, pour lesquels les mesures de restriction de l'activité sont extrêmement handicapantes. Or, nous le savons- et l'ensemble des professionnels de la montagne ont travaillé dans ce sens -, les mesures sanitaires peuvent et doivent être adaptées. Et nous devons continuer à vivre : oui, nous devons apprendre à vivre avec le virus Les acteurs de la montagne veulent travailler : laissez-les donc travailler ! Cette volonté est tellement forte qu'une petite station des Hautes-Alpes, Saint-Léger-les-Mélèzes, a décidé de pallier la fermeture des remontées mécaniques en utilisant un cheval de trait, afin d'enseigner le ski de piste aux plus jeunes. Que dire de plus ? Aussi, je dénonce de nouveau le manque total de visibilité, en particulier en ce qui concerne les vacances de février, période incontournable qui correspond à 40 % à 50 % du chiffre d'affaires pour nos stations et pour le tourisme hivernal. Le Premier ministre vient à l'instant de déclarer : « Je suis optimiste, mais cela demande confirmation. Je salue le comportement des Français pendant les fêtes. » Alors, monsieur le secrétaire d'État, quel est le calendrier gouvernemental pour les vacances de février ?

des périls économiques et sociaux auxquels font face les territoires de montagne, mais certains acteurs restent inéligibles à ces aides. Je pense plus particulièrement aux hébergeurs de montagne ou aux régies publiques de remontées mécaniques, généralement adossées à de petites communes, qui ne semblent pas, à ce jour, éligibles aux mesures de soutien. Je demande au Gouvernement d'accroître les aides financières en faveur de la montagne et d'élargir les critères d'éligibilité. Joël Giraud nous a annoncé, et je l'en remercie, une « logique valléenne » pour l'accompagnement territorial, mais j'ai aussi entendu

du maintien des populations rurales, de la biodiversité, des paysages, de l'aménagement du territoire et, bien entendu, du développement de l'économie touristique. Le maintien de montagnes vivantes passe inévitablement par le développement de l'activité économique. Or, dans certains territoires, notamment dans les Pyrénées, et particulièrement en Ariège, les éleveurs doivent faire face à la présence de prédateurs qui se livrent très régulièrement à des attaques de troupeaux. Ces attaques répétées des ours affectent dramatiquement le quotidien des éleveurs. Cette situation a pour conséquence directe de faire régresser le pastoralisme, souvent par découragement. Les éleveurs transhumants aspirent à pouvoir exercer leur travail dans de bonnes conditions, sans pression extérieure d'un prédateur peu maîtrisé. Monsieur le secrétaire d'État, nous savons tous que l'ours est une espèce strictement protégée au titre de la convention de Berne et de la directive européenne Habitats-faune-flore. Mais cette convention date de 1979 : à cette époque, l'Europe comptait neuf membres et les ours slovènes étaient en voie de disparition. Aujourd'hui, l'Europe se compose de vingt-huit membres, et alors que la France s'escrime à introduire des ours slovènes à grands frais au risque de voir se réduire l'activité pastorale, la Slovénie abat de son côté plusieurs dizaines d'ours par an. Si vous avez quelques milliers d'euros à dépenser, vous pouvez aller tuer un ours en Slovénie quand, dans les Pyrénées, on s'évertue à grand renfort d'argent à maintenir cette même population slovène délocalisée. Vous le voyez, monsieur le secrétaire d'État, depuis 1979, les choses ont bien changé. Ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de demander aux instances européennes de rediscuter de cette directive et d'envisager la sauvegarde des espèces à l'échelon européen avec un budget dédié ?

pour évaluer la situation sur le terrain et formuler un certain nombre de recommandations, qui se sont traduites par une feuille de route adoptée en juin 2019 et actualisée en juin 2020. Celle-ci intègre désormais les orientations du Président de la République,

la réplique. Je suis bien conscient que la perception de nos concitoyens dépend du lieu dans lequel ils résident. En effet, plus on s'éloigne de la montagne, plus l'ours ressemble à la peluche de notre enfance ... Pourtant, l'ours est une bête dangereuse : faudra-t-il attendre des drames humains pour que des décisions énergiques et de bon sens soient prises ?

Monsieur le secrétaire d'État, je me demande si ce n'est pas vous qui avez donné le mauvais exemple dès le départ, en éveillant le goût pour la parole chez tous nos collègues ! Madame la présidente, puisque nous nous connaissons, vous savez bien que je donne souvent le mauvais exemple,

particulièrement sensible à la tenue de ce débat dans notre enceinte. Il y a peu, notre assemblée a déjà eu l'occasion de travailler sur ces questions, avec notamment le rapport d'information de notre collègue Cyril Pellevat, qui examinait l'application de la loi Montagne II.

Toutefois, il faut se projeter au-delà de cette crise et envisager un développement économique et humain durable de nos zones de montagne qui prenne en compte l'ensemble des changements en cours et qui préserve notre environnement. Nous avons déjà eu ici l'occasion d'évoquer la situation difficile de certaines filières, en en particulier celle du bois, compte tenu des difficultés parasitaires. Globalement, le changement climatique a d'ores et déjà un impact sur nos massifs montagneux. Il montre les limites d'un développement économique fondé en grande partie sur un tourisme de sports d'hiver de masse. Les collectivités territoriales et les élus de terrain, en coordination avec les acteurs économiques, tentent de mettre au point des stratégies alternatives centrées sur le tourisme « 4 saisons », mais aussi sur les activités culturelles, les richesses gastronomiques et culinaires, nos sites naturels et la variété de l'artisanat local.

qui ne sont pas toujours faciles à mettre en oeuvre en France- il faut bien le reconnaître -, parce que nous disposons rarement de filières complètement intégrées nous permettant un véritable développement- je pense en particulier à la filière bois. Pour autant, des expériences

À cette rareté du foncier s'ajoutent des phénomènes qui peuvent encore accroître la pression foncière. C'est le cas dans les stations de ski renommées ou encore les communes frontalières. Dans ces zones, le prix du mètre carré constructible peut atteindre 11 000 euros. Quand neuf logements construits sur dix sont devenus des résidences secondaires, c'est la population permanente de ces communes qui fuit et des stations qui se meurent. Ce sont des services publics, des entreprises, des hôpitaux, des Ehpad qui ne parviennent plus à recruter, des classes d'écoles qui ferment, tant le prix du logement et du foncier devient inabordable pour la grande majorité des citoyens. Face à cette situation, les élus sont démunis et ont bien peu de moyens pour enrayer ces phénomènes. À mon sens, nous sommes ici dans le cas où la différenciation et la reconnaissance de la spécificité des zones de montagne doivent pouvoir pleinement s'appliquer. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles : nous devons accorder aux élus locaux des moyens réglementaires pour les aider dans cette tâche. Certains maires, à l'instar d'Éric Fournier, maire de Chamonix, ont déjà pris des mesures courageuses. Relayant une proposition de Mme le maire de Megève, j'ai suggéré il y a quelques mois à Julien Denormandie, alors ministre du logement, de mettre en oeuvre une expérimentation visant à accorder dans ces communes un abattement significatif des droits de succession à tout héritier, en contrepartie de son engagement à s'établir durablement dans la commune au titre de sa résidence principale. Cette piste me paraît intéressante à creuser, mais ce n'est pas la seule : il faut également se pencher sur la problématique des zonages A, B, C affectés à de nombreuses communes, qui se révèlent inadaptés et qui les privent de nombreuses aides à l'investissement locatif intermédiaire.

qui sont relativement riches et proches des grandes agglomérations internationales- je pense en particulier au bassin économique de Genève -, avec des problèmes de spéculation immobilière et d'artificialisation de l'offre. Vous évoquez la pression foncière dans un certain nombre de stations et les pistes qui ont été trouvées à Megève ou à Chamonix, où les prix au mètre carré sont plus élevés qu'à Lyon. Je connais bien cette situation, qui n'est pas tout à fait la même dans tous les massifs la même attractivité, car tout le monde n'a pas Genève et l'aéroport de Cointrin à proximité immédiate. Les grandes capitales européennes du Nord sont toutefois très proches des Alpes, ce qui crée des situations difficiles. Ma réponse comporte deux volets principaux. D'abord, il existe une notion de zone tendue en montagne, comme il existe des zones de revitalisation rurale en montagne. Ces zonages fiscaux ne permettent pas toujours de rendre compte de la réalité de la tension du marché, j'en suis d'accord. Ce n'est d'ailleurs pas spécifique à la montagne. Des travaux sous l'égide d'Emmanuelle Wargon sont en

de l'urbanisme et de la cohésion des territoires, les PLUI et les SCOT sont évidemment des outils pertinents pour freiner la tension foncière. Certaines communes et intercommunalités ont pu innover avec succès : elles méritent d'ailleurs d'être reconnues et soutenues. La réponse à la question posée passe souvent par une stratégie territoriale à l'échelon intercommunal du SCOT, qui me semble constituer l'une des priorités.

un tissu économique qui se délite complètement face à cette fuite de population permanente. Les professionnels n'arrivent même plus à subvenir à leurs besoins en dehors des périodes touristiques. Il y a donc vraiment urgence à agir.

cette problématique. La parole est à M. Cédric Vial. Nous savons désormais que la crise sanitaire et les décisions politiques qui l'ont accompagnée feront des zones de montagne, dont beaucoup vivent de l'industrie du tourisme, les territoires les plus sinistrés de France. Il faut donc panser et réparer pour permettre à ces acteurs de survivre. Il faudra ensuite penser et investir pour permettre à ces habitants de continuer à pouvoir y vivre. Si je salue l'effort consenti par le Gouvernement dans le décret du 30 décembre, un certain nombre de situations restent encore à ce jour sans réponse. Je pense notamment aux agriculteurs pluriactifs, qui travaillent également comme saisonniers : moniteurs de ski, pisteurs ou dameurs. Disposant d'un seul code NAF, ils ne peuvent bénéficier d'aucune aide pour leur activité saisonnière. Or, sans la prise en compte de cette double activité, ils ne s'en sortiront pas. C'est donc une grande partie de notre agriculture de montagne qui risque de s'effondrer avec eux. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous rassurer sur la prise en compte de ces situations par le Gouvernement dans les meilleurs délais ? Je souhaite aussi appeler votre attention sur la situation des entreprises gérant plusieurs établissements, comme c'est le cas de nombreux restaurateurs, loueurs de matériel, mais aussi des résidences de tourisme ou des centres de vacances. Il apparaît nécessaire de transformer le plafond des aides prévues par entreprise en un plafond d'aide par établissement, dans la limite du plafond européen de 800 000 euros et, si possible, en permettant à certaines d'entre elles de déroger à ce plafond.

La fonte des capacités d'autofinancement que cette crise aura provoquée fait courir de gros risques de décrochage à des territoires entiers qui, avant cette crise, avaient les capacités et la volonté de faire face aux enjeux climatiques et à la nécessaire diversification sur laquelle s'appuie un grand pan de l'économie de montagne.

Malgré le dernier décret, nous constatons que le Fonds de solidarité n'est pas adapté. Si l'on ne veut pas la disparition et la destruction, en un seul trimestre, de ce modèle économique de plus de soixante ans, il est nécessaire de protéger mieux l'ensemble des acteurs. Tous les types de commerces - hébergeurs, résidences de tourisme, villages et centres de vacances, mais aussi médecins et pharmaciens, fournisseurs alimentaires ou de matériel - ont besoin d'une prise en charge de 70 % de leurs frais fixes sur une année, de décembre à décembre,

saison. Monsieur le secrétaire d'État, dans quel délai le Gouvernement entend-il prendre des mesures complémentaires de survie, afin que ne disparaisse pas l'économie de la montagne, générée directement ou indirectement par les stations en termes de ressources et d'emplois, que les nombreux investissements et efforts déjà réalisés dans le sens d'une montagne durable ne l'aient pas été en vain, et que, tout simplement, la vie même de toutes les familles concernées soit préservée ? La parole est

notamment en raison de son modèle économique, puisque les charges fixes, incompressibles, sont structurellement très élevées. Certes, les acteurs du secteur bénéficient des mesures de soutien aux entreprises mises en place par le Gouvernement,

face à la crise sanitaire et à l'absence de visibilité pour le redémarrage de leurs activités. Je souhaite aborder un autre sujet. Alors que nos communes de montagne disposent de nombreux atouts qui contribuent au rayonnement de notre pays, leur attractivité est aujourd'hui fortement pénalisée par l'absence de certains services de première nécessité, notamment un accès correct à la téléphonie mobile. Je pense ainsi à un médecin, forcée de quitter sa commune, car elle ne pouvait assurer ses gardes en temps de crise sanitaire, à des habitants vivant en contrebas d'un barrage, qui craignent de ne pouvoir être informés en cas de danger, à un maire obligé de dormir dans sa mairie mairie pour prendre connaissance des directives du Gouvernement durant le confinement. Ce fut et c'est encore le quotidien des habitants de plusieurs communes en Isère, comme ailleurs en France, notamment en secteur de montagne. C'est la raison pour laquelle j'aimerais attirer une nouvelle fois votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur les problèmes de réseau et les zones blanches de la téléphonie en montagne. Comme l'illustrent les exemples que je viens de citer, les habitants de ces communes ne peuvent ni communiquer, ni télétravailler, ni s'informer, ni s'instruire - je pense aux plus jeunes -, ni accéder aux services publics dématérialisés. Les conséquences sont aussi de nature économique. En station de ski, certains acteurs rencontrent des difficultés pour louer leur bien, souffrant ainsi d'un handicap par rapport aux territoires voisins. Cette situation engendre, dans ces communes de montagne, un sentiment de marginalisation. Alors que l'on débat du déploiement de la 5G dans nos métropoles, certains habitants n'ont toujours pas de connexion portable correcte ni même la 4G. En 2018, votre gouvernement a annoncé un nouveau programme, le « New Deal mobile », censé régler la question de la couverture mobile et de la 4G. Force

à ce jour du « New Deal mobile » dans les zones de montagne et, plus généralement, de l'inclusion numérique de ces communes ? Que comptez-vous faire pour accélérer le déploiement de la 4G dans ces zones et rattraper le retard ?

sites ont migré en 4G ces derniers mois. En zone de montagne, entre juin 2017 et 2020, 5 114 sites 4G ont été activés pour atteindre un total de 8 200 sites 4G

face à une incompréhension globale des acteurs, qui font pourtant tout pour s'adapter aux conditions sanitaires imposées par le virus. Ils ont mis en place un protocole totalement abouti et validé par les services de l'État, afin que les remontées mécaniques puissent rouvrir avec une sécurité sanitaire maximale.

Les chiffres du tourisme hivernal, qui ont été donnés par plusieurs de mes collègues, sont éloquents. Sans ouverture, ce ne sont pas uniquement les entreprises et les salariés qui en subiront les conséquences

Les conséquences d'une absence d'ouverture risquent d'être la destruction définitive et irréversible du modèle économique de la montagne. Nous risquons de le voir disparaître en l'espace d'un trimestre.

sont aussi des centaines de millions d'euros de recettes en moins pour le budget de ces communes. La réalité, ce sont les choix cornéliens que devront faire nos élus pour gérer au mieux leurs services publics locaux et répondre à un intérêt général en souffrance.

Nos territoires de montagne, qui sont essentiellement ruraux, pourraient ainsi être mieux soutenus. Je sais, monsieur le secrétaire d'État, que vous êtes vigilant sur ce dossier. Utiliser le vieux serpent de mer d'une réforme globale des finances pour rejeter cette évolution de justice montre à quel point les réalités rurales ne sont pas toujours écoutées.

des solutions à ce que l'on appelle un « handicap naturel », il convient d'améliorer les communications terrestres, aériennes et numériques. Garder nos territoires accessibles et les laisser ouverts sur les autres est une condition essentielle de leur développement ou plutôt, à l'heure actuelle, de leur survie.

Il est également primordial que la rénovation du réseau ferré devienne une réalité. Le Président de la République a lui-même affirmé qu'il fallait développer massivement

La montagne, c'est aussi un art de vivre. La crise sanitaire nous enseigne que les citadins aspirent à un retour à la nature, à l'espace et à la montagne.

qui lie la quiétude et la solitude des grands espaces à des activités économiques vitales telles que l'agriculture et le tourisme. Monsieur le secrétaire d'État, nous comptons sur vous pour valoriser ce patrimoine et soutenir toutes les activités montagnardes et leurs potentiels.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, présentée par MM. Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte, Hervé Maurey et plusieurs de leurs collègues

je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cet hémicycle pour tout d'abord nous souhaiter une très bonne année 2021 et pour examiner la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France.

Il s'appuie sur les travaux que nous avons menés, à savoir des auditions, des contributions et des concertations avec tous les acteurs concernés, mais aussi avec le Gouvernement, ou encore une étude chiffrée inédite et prospective sur l'évolution de l'empreinte carbone du numérique en France. l'heure est donc à la concrétisation et à l'aboutissement de cet important travail précurseur que nous avons su engager au Sénat. Monsieur le secrétaire d'État, vous ne serez donc pas étonné que je commence par vous solliciter pour nous assurer de l'avenir de ce texte, dans le cadre de la navette parlementaire. Je connais votre engagement sur ce sujet et je sais que vous en partagez l'objectif. À l'origine de notre démarche, il y avait un constat et un objectif. Le constat, c'est que le numérique et ses usages explosent en France comme partout dans le monde. Les périodes inédites de confinement que nous avons vécues sont d'ailleurs venues fort à propos nous rappeler à quel point nous en avons besoin. Ce développement est indispensable à la transition écologique, notamment par les innovations qu'il permet dans les secteurs industriels les plus polluants. ces gains sont associés à des impacts directs et quantifiables en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation des ressources halieutiques, de consommation d'énergie et d'utilisation d'eau douce. Notre objectif était donc clair : agir sans attendre, prendre le tournant de la transition numérique, tout en s'assurant que ce secteur indispensable à la transition écologique ne devienne pas une source de pollution exponentielle. C'est justement parce que nous croyons à l'importance et à la nécessité du numérique que nous souhaitons l'inscrire sur la trajectoire responsable qui nous permettra de respecter nos engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris. J'entends certaines interrogations qui ont été formulées. Pourquoi une régulation climatique pour ce secteur plutôt que pour un autre ? Parce que sa croissance et, donc, son empreinte environnementale explosent. Le numérique, c'est 2 % de notre empreinte carbone aujourd'hui, mais, potentiellement, près de 7 % demain si l'on ne fait rien. En outre, si nous ne soutenons pas dès aujourd'hui les filières de reconditionnement des terminaux numériques ou des centres de données énergétiquement sobres, d'autres le feront pour nous et nous serons dépassés. Vous me permettrez d'exprimer ma satisfaction de voir se concrétiser une initiative parlementaire doublement inédite.

inédite, car nous nous apprêtons à discuter une proposition de loi qui aborde pour la première fois les impacts environnementaux de l'ensemble de la chaîne de valeur numérique, des terminaux aux centres de données, en passant par les réseaux. Monsieur le secrétaire d'État, depuis que nous avons rendu publics, en juin, notre rapport et notre feuille de route, avec ses 25 propositions pour une transition numérique écologique, d'autres acteurs se sont penchés sur le sujet, et c'est tant mieux. le Conseil national du numérique a publié sa feuille de route en juillet. Vous-même vous êtes également saisi du sujet, notamment dans le cadre d'une feuille de route présentée conjointement avec votre collègue chargée de la transition écologique. Nous nous en réjouissons, mais nous pensons qu'il est temps d'avancer plus vite et d'aller plus loin. Nous proposons donc d'agir concrètement. Avant de présenter plus en détail le contenu de la proposition de loi, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'avis du Haut Conseil pour le climat sur l'impact environnemental du déploiement de la 5G, remis au président du Sénat le 18 décembre

de rappeler la genèse de l'avis important du Haut Conseil pour le climat. Le Sénat a pris ses responsabilités, sur proposition de la commission de l'aménagement du territoire

Il n'est pas surprenant que cet avis préconise une évaluation systématique de toute nouvelle technologie, précisément pour pouvoir avoir des débats éclairés sur des sujets si importants et non pas des oppositions stériles ou non documentées. documentées. Par ailleurs, sur le fond, cet avis conforte les conclusions de nos travaux. La 5G pourrait très largement contribuer à l'augmentation de 60 % de l'empreinte carbone du numérique en France d'ici à 2030. Dans son scénario « haut le HCC estime que la 5G pourrait conduire à elle seule à une hausse de 45 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur d'ici à 2030. La moitié de cet impact carbone serait liée au renouvellement ou à l'acquisition des terminaux. Si le Haut Conseil estime que la feuille de route gouvernementale n'apporte pas pour le moment de garanties, la somme des mesures proposées ne se traduisant pas par moins d'émissions, notre proposition de loi offre de nombreuses réponses aux recommandations formulées dans son avis. Il ne s'agit pas d'être anti-5G ! Il faut simplement accompagner le secteur pour prévenir les impacts induits par son déploiement. Dans le détail, les leviers d'actions identifiés par la proposition de loi sont au nombre de

d'une formation à ce que vous avez justement appelé, monsieur le secrétaire d'État, l'« écologie du code ». La mise à disposition, pour tous, d'informations fiables et objectives, la création d'observatoires de recherche des impacts environnementaux du numérique, est plébiscitée par tous les acteurs que nous avons entendus, ainsi que des outils permettant aux entreprises de prendre conscience de leur impact et de déployer des actions à même de les réduire. Le deuxième de ces leviers vise à limiter le renouvellement des terminaux, principaux responsables aujourd'hui de l'empreinte carbone du numérique. est l'objet du chapitre II, qui entend notamment lutter contre l'obsolescence programmée des logiciels, mais aussi contre ce que l'on pourrait appeler l'« obsolescence marketing », qui introduit un biais en faveur d'un renouvellement trop rapide des smartphones. Le chapitre III de la proposition de loi vise à promouvoir le développement d'usages du numérique écologiquement vertueux. La création d'un référentiel général de l'écoconception, auquel devront se conformer les plus grands fournisseurs de contenus, nous semble indispensable. Il est aujourd'hui possible de faire des sites aussi performants avec une quantité de données et, donc, d'énergie utilisée bien moindres. Enfin, le chapitre IV tend à la création de centres de données et de réseaux moins énergivores,

Une piste similaire est également envisagée par le rapport du Haut Conseil pour le climat. Je laisserai bien sûr le soin aux deux rapporteurs et à la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, que je salue, de présenter les nombreux apports adoptés en commission. Je me réjouis que le texte ait été enrichi d'un volet relatif à la promotion d'une stratégie numérique responsable dans les territoires. Pour ma part, nous y reviendrons lors de l'examen des articles, je vous proposerai un amendement tendant à ce que les biens reconditionnés ne soient pas soumis à une rémunération pour copie privée, dès lors que les produits ont déjà fait l'objet d'une mise sur le marché en Europe et ont déjà, à ce titre, été assujettis à ce prélèvement. Je proposerai également de compléter le chapitre de la proposition de loi relatif aux impacts environnementaux des réseaux. Il me paraît en effet important de lutter contre les pratiques spéculatives qui sont celles de certaines, engendrant des gels de terrains et, parfois, la construction d'infrastructures mobiles sans fourniture de services. Ces pratiques peuvent conduire à l'érection de pylônes inactifs, générant un impact environnemental inutile, par exemple une artificialisation des terres concernées. Voilà, mes chers collègues, les principaux points que je voulais vous présenter concernant cette proposition de loi que je vous invite bien sûr à adopter, et à laquelle je souhaite de connaître une navette fructueuse.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je suis très heureux de vous présenter, avec mon collègue corapporteur, la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, telle que modifiée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Avant d'entrer dans le détail de son contenu, je voudrais remercier, tout d'abord, les anciens membres de la mission d'information, mais aussi tous nos collègues de la commission qui, quel que soit leur groupe politique, contribué à enrichir ce texte, dans un état d'esprit rigoureux et constructif- c'est là la marque de fabrique du Sénat. Ce moment est important, car nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là, beaucoup écouté, et exploré de nombreuses pistes. C'est, au fond, la preuve que nos travaux de contrôle parlementaire peuvent jouer un rôle de vigie et d'impulsion très important pour la fabrique de la loi. J'en viens au contenu de la proposition de loi. Le premier axe vise à faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact environnemental. L'idée est de toucher tous les citoyens, les acteurs publics et les entreprises, afin de développer une « culture de la sobriété numérique L'article 1 fait de la sensibilisation à l'empreinte environnementale du numérique l'un des thèmes de la formation à l'utilisation responsable des outils numériques à l'école. L'article 2 généralise les modules relatifs à l'écoconception des services numériques dans les formations des ingénieurs en informatique, afin de permettre l'émergence de ce que l'on pourrait appeler une « écologie du code » dans ce secteur professionnel. L'article 3 crée un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique, placé auprès de l'Ademe, l'Agence de la transition écologique, pour analyser et quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement, ainsi que sa contribution à la transition écologique. L'article 4 prévoit d'inscrire l'impact environnemental du numérique dans le bilan de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). L'article 5 crée un crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises afin de les inciter, d'une part, à acquérir des équipements numériques reconditionnés et, d'autre part, à faire réaliser des études d'impact environnemental de leurs services numériques et, le cas échéant, à mettre en oeuvre une stratégie de transformation numérique durable de ces services. Le deuxième axe de la proposition de loi vise à limiter le renouvellement des terminaux, principaux responsables de l'empreinte carbone du numérique. À l'article 6, la commission a souhaité rendre plus opérant le délit d'obsolescence programmée, aujourd'hui concrètement inapplicable, en supprimant un des deux critères requis pour le caractériser. Je rappelle qu'aucune condamnation n'a été prononcée sur le fondement de ce délit depuis sa création en 2015.

en s'assurant que le consommateur soit informé, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour ; en augmentant de deux à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens ; en permettant à l'utilisateur ayant installé une mise à jour évolutive de rétablir les versions antérieures des logiciels. L'article 11 fait passer de deux à cinq ans la durée de la garantie légale de conformité pour les équipements numériques. L'article 12 prévoit que les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés

Pour en faire un levier d'accroissement de la durabilité des produits numériques, il prévoit la prise en compte de critères de durabilité des produits dans les achats publics de certains produits numériques. L'article 13 A, introduit en commission, vise à ce que la sobriété numérique et la durabilité des produits soient inscrites dans les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables des plus grandes collectivités territoriales. L'article 14 prévoit de réduire le taux de TVA sur la réparation de terminaux et l'acquisition d'objets électroniques reconditionnés pour limiter les achats neufs. Nous savons les difficultés de conformité au droit européen soulevées par cet article, mais nous souhaitons vous proposer que le Sénat exprime une position forte sur ce sujet, dans la perspective d'une éventuelle révision de la directive TVA au niveau européen. Enfin, la commission a souhaité mieux lutter contre l'obsolescence « marketing » en introduisant un article 14 qui renforce l'information du consommateur concernant les offres « subventionnées », qui, associant l'achat d'un smartphone à la souscription d'un forfait mobile, peuvent induire un biais en faveur du renouvellement

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je poursuis donc l'exposé de mon collègue par le troisième axe de la proposition de loi, qui appelle à faire émerger et à développer des usages du numérique écologiquement vertueux. L'article 15 prévoit que les opérateurs privilégient des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. L'article 16 crée une obligation d'écoconception des sites des plus gros fournisseurs de contenus, qui occupent aujourd'hui une part très importante de la bande passante. Ils devront se conformer à un référentiel général de l'écoconception, qui fixera notamment les règles relatives à l'ergonomie des services numériques, ainsi qu'à l'affichage et à la lecture des contenus multimédias. Les articles 18, 19 et 20, qui prévoyaient respectivement l'adaptation de la qualité des vidéos téléchargées à la résolution maximale du terminal utilisé, l'interdiction du lancement automatique de vidéos et l'interdiction du défilement infini, ont été satisfaits par les modifications ainsi apportées par la commission, et ont donc été supprimés. Le référentiel général de l'écoconception intégrera également des critères permettant de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs, afin de rendre plus opérationnelle la disposition initialement prévue à l'article 17, qui a lui aussi été supprimé. Les travaux engagés sur le référentiel portent déjà leurs fruits, puisque nous avons très récemment appris qu'un travail des services de l'État et de l'Ademe était en cours sur ce sujet dont traite l'article 16. J'en viens aux orientations du chapitre IV de la proposition de loi, visant à promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores. À l'article 21, la commission a souhaité réitérer la position exprimée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, en prévoyant que l'octroi du tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation à l'atteinte d'objectifs environnementaux pluriannuels ; elle considère en effet que le dispositif adopté dans le cadre du projet de loi de finances sur l'initiative de l'Assemblée nationale ne constituait pas une incitation fiscale réelle au verdissement des centres de données. L'article 21 , introduit en commission, permettra par ailleurs aux plus petits centres de données de bénéficier également de ce tarif réduit de TICFE, ce qui les incitera à s'engager eux aussi dans un tel verdissement. L'article 22, pleinement satisfait par les modifications apportées à l'article 21, a été supprimé. À l'article 23, la proposition de loi prévoit que les opérateurs de réseaux souscrivent des engagements environnementaux pluriannuels contraignants, au plus tard en 2023. Dans ce cadre, les opérateurs devront aussi s'engager à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l'utilisation des box des box mises à disposition de leurs abonnés, et à planifier l'extinction progressive des anciennes générations de réseaux mobiles, toujours consommatrices d'électricité.

offrira un cadre de régulation pertinent, à l'heure où les consommations et les émissions des réseaux devraient augmenter avec le déploiement de la 5G, comme l'a rappelé le récent rapport du Haut Conseil pour le climat, auquel il a été fait allusion tout à l'heure. L'article 24 permettra l'inscription de critères environnementaux minimaux dans les licences mobiles attribuées par l'Arcep. Je note que le rapport du Haut Conseil pour le climat sur la 5G formule des propositions très proches à l'article 23 , introduit en commission, il permettra à l'Arcep de récolter les données qui lui seront nécessaires pour assurer cette régulation. La commission a en outre souhaité compléter la proposition de loi par un chapitre relatif à la promotion de stratégies numériques responsables sur les territoires. L'article 25 prévoit que les plans climat-air-énergie territoriaux programment des actions visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique et intègrent le potentiel de récupération de chaleur des centres de données dans leur stratégie. L'article 26 prévoit l'élaboration par les plus grandes collectivités d'une stratégie numérique responsable, présentée chaque année en amont du débat budgétaire. Voilà, mes chers collègues, les grandes lignes de cette proposition de loi, que nous avons voulue ambitieuse et équilibrée. À mon tour, je souhaite remercier nos collègues de la commission de l'aménagement du territoire et de la commission des affaires économiques, avec qui nous avons travaillé en bonne intelligence tout au long de cet examen. Ce texte est important, comme le montrent la mobilisation et la forte implication de toutes les sensibilités de notre hémicycle. Monsieur le secrétaire d'État, j'espère que vous pousserez cette initiative, qui mérite que nous travaillions de concert. Je vous souhaite à tous une bonne année numérique responsable

avis. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer le travail de mes collègues Patrick Chaize, Hervé Maurey, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte et à les remercier pour leur écoute et pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans nos échanges. Cette proposition de loi permet au Sénat d'aborder, en précurseur, la question de l'empreinte environnementale du numérique. Elle vient compléter la loi sur l'économie circulaire, un an après sa publication et alors que nombre de ses dispositions, comme celle sur l'indice de réparabilité, entrent tout juste en vigueur en ce début d'année. Si l'impact environnemental du numérique apparaît à ce jour relativement limité en France, l'explosion prévisible des usages devrait l'aggraver dans les décennies à venir- cela a été dit. Pour autant, nous ne disposons pas de chiffrage des émissions « évitées par le recours grandissant au numérique. L'approche coûts-avantages du numérique reste donc à consolider au fur et à mesure des développements des usages et au regard des estimations disponibles, celle de la Commission européenne notamment, qui font état d'une réduction des émissions égale à sept fois les émissions générées par le numérique lui-même. Le numérique est indéniablement un levier majeur de la transition écologique, mais il est vrai que ses modalités de déploiement restent à parfaire afin de mieux maîtriser nos impacts environnementaux et d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est ce qui est visé dans cette PPL : appliquer la transition écologique à la transition numérique. Pour atteindre cet objectif de soutenabilité du numérique, il s'agit de mettre en place et de diffuser des pratiques plus vertueuses, chez l'ensemble des acteurs : fabricants de terminaux et d'équipements, concepteurs de logiciels et d'applications, distributeurs, opérateurs, mais aussi usagers. La singularité de cette proposition de loi est précisément de s'intéresser à l'ensemble des acteurs de cette chaîne, et aux particularités de chacun. de chacun. Pour réduire notre empreinte numérique, c'est-à-dire l'impact environnemental de notre consommation numérique, l'une des priorités doit être l'allongement de la durée de vie des terminaux que nous utilisons : ordinateurs, téléphones, écrans, télévisions. Cet enjeu majeur repose à la fois sur les fabricants, mais aussi sur nous, consommateurs, qui devons nous défaire de cette course effrénée au « dernier modèle sorti ». Concernant la fabrication de ces équipements, l'empreinte environnementale est principalement liée aux importations, une fois encore. La France devra donc, au-delà de cette PPL, porter une stratégie à l'échelle européenne et internationale. Mais tout commence avec ses propres engagements ; ce texte vise donc à fixer un cadre et à engager sans tarder les acteurs domestiques français dans la transition écologique. La commission des affaires économiques a cherché, dans cette première phase de transition, à privilégier l'incitation. Cela nous est apparu essentiel dans le contexte de grandes tensions économiques que nous abordons accélérer la transition écologique sans négliger les surcoûts qu'elle engendre pour les ménages comme pour les entreprises. Comme nous l'avons proposé pour les, il nous semble nécessaire d'inciter en suscitant leur adhésion et en créant des conditions économiques attractives et une véritable dynamique de changement, en définitive plus vertueuse, car lesdits acteurs y souscrivent plus rapidement et en nombre, tout en minimisant les distorsions de concurrence que créent nécessairement les systèmes contraignants franco-français. Tout au long de l'examen de ce texte, nous avons donc privilégié autant que possible une écologie incitative, fondée dans un premier temps sur des accompagnements fiscaux, ceux-ci étant destinés à évoluer, voire à disparaître au fur et à mesure de la mise en oeuvre des directives européennes convergentes en oeuvre des directives européennes convergentes qui seront prises dans les mois à venir. Cette démarche s'inscrit dans l'approche européenne de régulation du numérique qui s'écrit depuis quelques mois et qui est d'actualité ces derniers jours celle du retour des États et d'une gouvernance partagée du numérique, une corégulation tripartite associant État, usagers et acteurs économiques, chacun ayant une responsabilité identifiée. Avec ce texte issu des travaux des commissions, nous parvenons à esquisser cette délicate ligne de crête. Le texte fixe à 2023 l'entrée en vigueur des dispositions lorsqu'il est nécessaire de disposer au préalable de méthodes standardisées et de données incontestables permettant d'établir des référentiels. Il proportionne la contrainte aux enjeux- je pense notamment à l'article sur l'écoconception des services en ligne, qui est ciblé sur les acteurs qui consomment le plus de bande passante dans les réseaux. Il incite, autant que possible, les acteurs économiques à s'engager dans une transition écologique vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour la compétitivité des entreprises établies établies en France- je pense notamment aux articles sur les. La commission des affaires économiques aurait préféré que l'incitation soit également préférée à la contrainte pour les opérateurs télécoms. Par ailleurs, afin de responsabiliser les utilisateurs plutôt que de les pénaliser, la proposition de loi leur redonne du pouvoir de décision, instaurant davantage de transparence en matière de mises à jour logicielles. Enfin, le texte issu des travaux de nos commissions est juridiquement consolidé face à un droit européen contraignant. contraignant. La commission des affaires économiques a appréhendé cette proposition de loi préfiguratrice d'un nouvel ordre numérique avec pour maîtres-mots « responsabilisation », « transparence » et « incitation ». La parole Madame la présidente, madame, messieurs les rapporteurs, monsieur le sénateur Chaize, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis ravi d'être parmi vous, en cette fin de journée, afin de débattre d'un sujet qui est- nous en sommes d'accord -très important, celui de l'empreinte environnementale du numérique. La mission d'information menée par les sénateurs Chaize, Chevrollier et Houllegatte a approfondi cette question au début de l'année dernière, aboutissant aujourd'hui à la proposition de loi que nous examinons. Je sais que nombre d'entre vous, au-delà de cette mission, se sont emparés de ce sujet, notamment les sénateurs Maurey et Loisier, et je tiens à saluer la qualité des travaux qui ont été produits à cette occasion. Ils s'inscrivent dans une riche dynamique, à la fois intellectuelle et opérationnelle- ont été cités la Convention citoyenne pour le climat, le Conseil national du numérique, appuyé par le Haut Conseil pour le climat, le récent rapport de l'Arcep ou divers travaux de collectifs et think-tanks,

Dans la famille politique dont je suis issu, la gauche, le progrès a d'ailleurs été historiquement une condition de l'émancipation. Je crois que cette vérité demeure, mais également que l'ADN de la France est d'assumer ce chemin vers la modernité. Ceux qui voudraient revenir aux formes anciennes du monde oublient, par idéologie, parfois par manipulation, que c'est bien le progrès, scientifique, technique, technologique, qui nous a permis de guérir, de prospérer, de réduire les inégalités, bref, de mieux vivre que quand la France a été tentée par une forme de conservatisme, de retour à une terre qui « ne ment pas », c'était toujours dans les périodes les plus noires de son histoire. Mais je crois aussi- et je crois que nous partageons cette préoccupation -que l'innovation n'est pas bonne en soi,

Lorsque se jouent des sujets aussi importants que ceux de l'avenir technologique de notre pays et aussi- ne l'oublions pas -de son avenir économique, à la croisée de questionnements environnementaux, alors il est de la responsabilité du politique de ne pas rester à la surface des choses. Je remarque, du reste, que c'est ce qui se passe, par exemple, dans le débat sur la 5G : les réticences s'amenuisent à mesure que le débat va au fond des choses, interrogeant la réalité des sujets sanitaires ou environnementaux. Je crois enfin que le progrès doit être mis au service d'une cause profonde et ontologique, celle de la préservation de l'environnement, absolument décisive pour le présent et pour l'avenir. Je crois même que cette relation entre numérique et environnement est plus profonde encore qu'il n'y paraît : la transition écologique, notamment la transition énergétique, ne sera possible qu'avec le numérique, pour une raison simple qui touche à l'essence même de la transition environnementale. Celle-ci repose très largement, en effet, sur un problème mathématique d'optimisation des ressources sous contrainte, s'agissant de ressources limitées. Elle repose aussi sur des fonctionnements beaucoup moins centralisés et beaucoup plus répartis- c'est le cas par exemple des ou encore des circuits courts. Or optimiser à grande échelle et en temps réel une répartition des ressources ainsi construite, particulièrement dans un contexte de pénurie, est un problème insoluble pour l'esprit humain- c'est d'ailleurs ce que montre extrêmement bien Jean-Marc Jancovici, le président de. Un tel problème Un tel problème ne peut donc être résolu que par des réseaux très performants, une très forte connexion des acteurs et une utilisation intensive de l'intelligence artificielle. C'est notamment pour cette raison que nous avons besoin de nouveaux réseaux ; c'est notamment pour cette raison que nous avons besoin de la 5G. C'est pourquoi les avantages de ces technologies, leurs gains écologiques embarqués, sont probablement bien supérieurs à leur consommation propre.

nous avons besoin de beaucoup plus d'innovation pour soutenir le défi environnemental, et pas de beaucoup moins d'innovation ! C'est cette responsabilité qui est la nôtre, et c'est cette responsabilité qui, d'ailleurs, irrigue le plan de relance qui a été porté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. Par la mobilisation inédite qu'il institue, nous accélérons concrètement le verdissement de l'économie tout en promouvant l'innovation et la compétitivité. C'est d'ailleurs, pour en revenir au texte de cette proposition de loi, de cette responsabilité qu'il s'agit ce soir. soir. Si, comme je viens de le dire, le numérique est globalement très favorable à la transition écologique, et particulièrement à la transition énergétique, cela ne l'exonère bien évidemment pas de porter sa part des efforts de sobriété et surtout d'efficacité qui sont nécessaires. ce sens, la volonté qui anime votre proposition de loi rejoint celle du Gouvernement telle qu'elle s'exprime dans le cadre de sa feuille de route interministérielle visant à faire converger numérique et écologie, que j'aurai l'occasion de présenter début février avec Barbara Pompili. Permettez-moi de revenir en détail sur les premiers axes de cette feuille de route que nous avons lancée en octobre dernier. Nous voulons tout d'abord objectiver l'empreinte environnementale du numérique et développer la connaissance que nous avons de ce sujet : mieux connaître pour mieux agir, en quelque sorte. perspective, nous avons confié à l'Ademe et à l'Arcep la mission de mener une étude approfondie visant, d'une part, à objectiver l'empreinte environnementale des réseaux de télécommunication fixe et mobile en fonction des usages qu'ils supportent et, d'autre part, à proposer des mesures de maîtrise et de réduction de leur impact, par exemple le démantèlement des réseaux anciens et redondants. Cette mission est évidemment importante pour la suite de nos échanges sur votre proposition de loi. Nous souhaitons, deuxièmement, faire du numérique un levier majeur de la transition écologique- j'ai eu l'occasion de le dire. Le numérique est en effet aujourd'hui une condition indispensable de la transition environnementale sans numérique, pas de voiture électrique ; sans numérique, pas de réseaux intelligents et pas de massification des énergies renouvelables ; sans numérique, pas d'agriculture de demain, plus économe en consommation de ressources et de produits phytosanitaires ; sans numérique, pas de transports ni de logistique optimisés, donc moins consommateurs d'énergie sans numérique, enfin, pas de gains de productivité indispensables à l'acceptabilité sociale de la transition environnementale. C'est pourquoi, dans le cadre du plan de relance, un fonds de 300 millions d'euros destiné aux projets des start-up de l'environnement a été créé. Enfin, je l'ai dit, pour être globalement positif pour l'environnement, le numérique n'en doit pas moins prendre sa part dans la maîtrise de notre empreinte énergétique. Pour le dire plus clairement : oui, nous devons entrer dans une phase déterminée de maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique- c'est notre troisième axe. cette empreinte en agissant sur chaque étape du cycle de vie des équipements, en amont de la production, au niveau de l'usage et en aval, là où la fin d'une vie peut devenir le début d'une nouvelle. La Convention citoyenne pour le climat- cela a été dit -a voté de nombreuses propositions en la matière. Notre feuille de route comprend des actions visant à produire moins et mieux : réparabilité, reconditionnement, réemploi, écoconception. D'ailleurs, la mise en oeuvre de ces actions créatrices d'emplois localisés constitue également un enjeu de filière industrielle et d'emploi pour la France. En matière d'allongement de la durée de vie, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) a déjà prévu des avancées fortes- je le rappelle -, notamment l'indice de réparabilité ou l'extension de la garantie légale de conformité de six mois lorsque l'appareil subit une réparation dans les deux ans. Ce que nous souhaitons, c'est accélérer sur le reconditionnement de ces téléphones. Trop souvent- vous l'avez dit -, les reconditionneurs se heurtent aux politiques restrictives des fabricants de téléphones en matière de pièces détachées. C'est pourquoi la loi AGEC a prévu un encadrement du temps de mise à disposition desdites pièces.

Nous voulons par ailleurs inciter beaucoup plus au réemploi des plus de 100 millions de smartphones qui dorment dans les tiroirs des Français. Nous avons en ce sens engagé une concertation avec les opérateurs télécoms et les acteurs du reconditionnement en France.

afin d'identifier dans le détail les principaux postes de consommation et de définir des pistes de rationalisation. Vous le voyez, de nombreuses mesures rejoignent les préoccupations des auteurs de cette proposition de loi et les dispositions qui y sont promues. Comme Comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous abordons l'examen de ce texte de manière ouverte, même s'il s'agira de l'affiner au cours de la navette parlementaire- nous avons eu l'occasion d'en discuter. Nous sommes, à ce titre, largement favorables aux dispositions visant à faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de leur impact environnemental.

calendrier. Des textes, notamment, sont en cours d'élaboration ; je pense à la transposition des directives européennes 2019/770 et 2019/771 respectivement relatives aux contrats de fourniture de contenus et de services numériques et aux contrats de vente de biens,

Des concertations sont par ailleurs en cours avec les opérateurs télécoms et avec les plateformes ; elles seront conclues dans les mois à venir. Avec les opérateurs télécoms, qui sont concernés par plusieurs articles, nous avons ouvert une concertation approfondie sur des enjeux aussi essentiels que le reconditionnement, le renouvellement des terminaux ou la tarification des données. Ce sont des enjeux auxquels ils souscrivent déjà de façon volontaire et pour lesquels ils sont prêts à prendre des engagements inscrits dans la feuille de route sur le numérique et l'environnement, que j'ai annoncée Faire entrer ces sujets dans le champ de la régulation, comme le souhaitent les auteurs de cette proposition de loi, est un choix politique fort, mais sensible. C'est un nouveau cadre à construire, y compris à l'aune des pratiques et de la régulation européenne. Nous souhaitons donc continuer à débattre afin d'aboutir à des solutions dans le courant de la discussion. Notre position sur vos propositions en la matière traduit ainsi notre volonté d'avancer avec les opérateurs, en bonne intelligence. Nous partageons la volonté d'inscrire le numérique dans le grand mouvement et la grande obligation de la transition environnementale, en l'aidant à prendre sa juste part dans l'effort. Face aux grands acteurs du numérique dont l'actualité souligne bien la puissance, certaines actions ne pourront être efficacement menées qu'à l'échelle européenne.

Faire converger le numérique et la transition écologique, ce n'est pas une mode, c'est un impératif ! Les périodes de confinement que nous avons vécues ont montré avec acuité la convergence entre ces deux mouvements de fond, le numérique et l'écologie. Tous deux ont connu un saut le numérique, comme pilier de la société, et l'écologie, comme fondement nécessaire à notre survie et à celle de la nature. À nous de faire du premier le remède du second ! La parole

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes en janvier 2021, c'est l'occasion pour moi de nous souhaiter collectivement une bonne année ! C'est une évidence, le numérique est plus qu'omniprésent dans notre quotidien. Nous savons qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Après plus de vingt ans de croissance ininterrompue, il occupe une place prépondérante dans notre quotidien personnel et professionnel, et touche tous les citoyens. Nul besoin d'être un pour en faire l'expérience chaque jour. Car, comme l'affirmait le philosophe Michel Serres en 2010, « nous vivons un changement de monde ». Oui, en quelques années, notre quotidien a plus changé qu'au cours du siècle précédent. Et le rythme des évolutions s'accélère. Cela n'est pas sans engendrer, notamment, des problèmes d'adaptation dans la vie de tous les jours. Avec le téléphone « intelligent », ou smartphone, chacun dispose désormais dans sa poche d'une puissance considérable, d'un ordinateur nomade qui nous relie au monde en permanence et qu'il convient de réguler. L'attaque portée- n'ayons pas peur des mots -contre la démocratie américaine sur l'initiative de Donald Trump, utilisateur compulsif de smartphone s'il en est, est sans conteste l'illustration de ces dérives, qui appellent des réponses collectives fortes. Fort heureusement, le numérique n'est pas que cela. On lui doit la complète mutation de notre façon d'aborder le quotidien. Comme certains l'ont souligné avant moi, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons est un accélérateur qui, bien évidemment, nous interpelle au regard de la démultiplication des usages, mais pas En 2040, si tous les autres secteurs réalisent des économies de carbone, conformément aux engagements de l'accord de Paris et si aucune politique publique de sobriété numérique n'est déployée, le numérique pourrait atteindre près de 7 % des émissions de gaz à effet de serre de la France, un niveau bien supérieur à celui actuellement émis par le transport aérien. Cette croissance serait notamment portée par l'essor de l'internet des objets et les émissions des. Ce constat n'est pas celui d'une quelconque Cassandre de l'environnement, mais celui de la mission d'information mise en place sur l'initiative de notre collègue Patrick Chaize, et dont le rapport adopté en juin 2020 a débouché sur la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Oui, la question de l'empreinte environnementale du numérique dans notre pays est aujourd'hui un sujet de société sur lequel il est de temps d'arrêter une stratégie partagée. Mais, disons-le d'emblée, cette proposition de loi n'est en rien le procès du numérique et le fruit de réflexions de sénateurs « hors-sol » : bien au contraire ! D'ailleurs, les acteurs du numérique, à part peut-être certains représentants de ce qu'on appelle communément les GAFA, l'ont parfaitement compris. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de nombreux travaux sur le sujet comme le rapport du Conseil national du numérique, les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, le dernier rapport de l'Arcep, ou bien encore les initiatives d'experts ou de collectifs engagés. Cette proposition de loi, monsieur le secrétaire d'État, est en phase, vous l'avez dit le 2 décembre dernier lors de votre audition, avec la feuille de route que vous portez, car, comme vous nous l'avez indiqué, « il n'y aura pas de transition environnementale sans transition numérique ». À l'heure où la relance de l'économie, après la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons, doit plus que jamais être verte, il convient de dire sans ambiguïté aucune que les politiques publiques doivent s'appuyer sur les outils numériques afin d'accélérer et d'optimiser la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. C'est un fait acquis que le numérique facilite d'abord la mesure et le suivi des impacts environnementaux, et donc favorise une utilisation plus raisonnée des ressources naturelles. Il participe également de l'efficacité énergétique, induit une réduction des déplacements ou contribue à l'émergence de modèles économiques fondés sur les principes de l'économie circulaire. Le numérique doit ainsi être mis au service de la transition écologique. Cela passera notamment par l'exploitation des données environnementales ou par la mobilisation des technologies au service de la transition environnementale. Ces éléments sont essentiels afin d'assurer la convergence des transitions numérique et écologique. Il n'y aura pas de transition écologique sans transition numérique, mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Le secteur doit travailler sur sa propre empreinte environnementale. Les tendances sont incontestables, et l'une des principales vertus des travaux de la mission d'information et de cette proposition de loi est de mettre l'église du numérique au centre du village, donnant ainsi le « top départ » d'une stratégie devant mobiliser toutes les énergies. Dans le monde, comme en France, cela a été dit et redit, le numérique constitue une source importante de gaz à effet de serre. Il a également un impact sur l'épuisement des ressources naturelles, ainsi que sur la pollution de l'eau, de l'air et du sol. Malgré les efforts considérables des acteurs du secteur, l'accélération de la transition numérique entraînera nécessairement une augmentation de ses impacts, augmentation qui ne pourra sans doute pas être compensée entièrement par l'amélioration de l'efficacité énergétique du numérique. Ces impacts sont majoritairement liés aux terminaux, notamment à leur fabrication et à leur distribution. La question de l'empreinte environnementale du numérique est aujourd'hui centrale et ne se résume pas au seul totem de la 5G. Je suis de ceux qui, sans hésiter, affirment que la 5G n'est pas ce « grand Satan » que certains responsables, voyant sans doute là une martingale politique de court terme, dénoncent sans cesse et souvent de manière outrancière. Disons-le une fois pour toutes, la 5G est avant tout conçue pour servir les échanges de données de très haut débit relatifs à l'industrie, à la santé connectée et à la ville intelligente. Sans doute convient-il, monsieur le secrétaire d'État, d'expliquer, d'expliquer toujours et d'expliquer encore ce que cette nouvelle technologie a à offrir et en quoi elle participe de la transition environnementale, alors même que l'Europe vient de donner le coup d'envoi de son projet de recherche sur la 6G ! Cette parenthèse ouverte et refermée, nous ne pouvons que saluer les priorités mises en avant dans cette proposition de loi. Je pense particulièrement au volet éducatif, qu'il faut déployer, même s'il convient de dépasser le seul cadre des utilisations et de mettre en place une véritable sensibilisation citoyenne sur la question des usages et la façon dont on utilise physiquement l'appareil : choix d'un matériel réparable, question du suréquipement, utilisation d'équipements reconditionnés, bref, toute la chaîne de vie du matériel numérique. Limiter le renouvellement des terminaux, faire émerger des usages du numérique écologiquement vertueux, aller vers des centres de données moins énergivores et promouvoir une stratégie numérique responsable sur les territoires sont autant de sujets

L'examen du texte en commission nous a collectivement permis de dépasser certains écueils. La discussion nous permettra d'aller plus loin. Au final, chacun s'accordera pour dire qu'avec ce texte le Sénat fait oeuvre utile. Pour toutes ces raisons, nous voterons cette proposition de loi. La parole est à M.

nous examinons aujourd'hui cette proposition de loi transpartisane qui nous permettra, je l'espère, de compléter notre arsenal législatif pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris en 2015. Ces objectifs, en matière de numérique responsable, sont ambitieux : le Gouvernement vise zéro émission net de gaz à effet de serre et 100 % de biens et services numériques écoconçus d'ici à 2030. Pour l'heure, le numérique serait responsable de 2 % des émissions de gaz à effet de serre en France, soit 15 millions de tonnes d'équivalent carbone en 2019, avec une croissance de l'empreinte énergétique de 9 % par an. an. C'est bien cette croissance qui inquiète puisque, selon les projections, le numérique représentera 7 % du total des émissions en 2040 dans notre pays. Il apparaît donc indispensable d'agir au plus vite, au-delà des dispositions de la loi AGEC, sur la réparation et le réemploi pour que les gains environnementaux permis par le numérique ne soient pas annulés par ses impacts en termes de pollution et de consommation de ressources et de matières premières. À ce titre, la mission d'information sénatoriale pour une transition numérique écologique, qui a préfiguré la rédaction de cette proposition de loi, a permis de fournir des éléments concrets sur un sujet qui manquait de données. On a ainsi pu confirmer que 81 % de l'empreinte environnementale du numérique reposait sur le renouvellement des terminaux, notamment sur leur fabrication. C'est donc sur ce point que les efforts doivent être engagés en priorité, d'autant que près de 95 % des Français possèdent un portable. Les mesures contenues dans cette proposition de loi tendent à renforcer le rôle du consommateur- public ou privé -en visant notamment à mieux lutter contre l'obsolescence programmée et à augmenter la durée de vie des appareils, deux sujets qui concourent au rachat trop fréquent de terminaux. Nous vous proposerons des amendements afin de limiter le renouvellement des terminaux en encourageant les biens issus de l'économie de fonctionnalité, ainsi que les produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Les consommateurs, par des usages écologiquement vertueux du numérique, par des exigences croissantes et des achats responsables, entraîneront des changements durables dans les méthodes de conception. Nous sommes donc parfaitement en accord avec les dispositions de cette proposition de loi sur la formation des élèves à l'utilisation responsable des outils numériques, ainsi qu'avec l'inscription de l'impact environnemental des biens et services numériques dans le bilan RSE des grandes entreprises. À ce sujet, le récent rapport du Haut Conseil pour le climat est venu confirmer les craintes grandissantes relatives au déploiement de la 5G et son impact sur les émissions de CO2, en raison du renouvellement des infrastructures, des terminaux et de l'accroissement prévisible des usages. Bien sûr, il ne s'agit pas de brider le numérique, mais il s'agit de rappeler que ce secteur ne doit pas être exempté d'efforts pour respecter les engagements climatiques de la France. Ce secteur comprend aussi bien les acteurs économiques, les consommateurs que les acteurs publics. Nous devons tous prendre notre part dans le déploiement d'un numérique responsable et vertueux. Cette proposition de loi offre une initiative législative complète en appréhendant toute la chaîne de valeur numérique. Il paraît donc important de rappeler que les collectivités et l'État aussi peuvent et doivent être moteurs et exemplaires en la matière. Cela passe par la commande publique, comme le prévoit l'article 13, qui vise à rendre obligatoire le recours aux produits numériques dont les critères de réparabilité, dans un premier temps, et de durabilité, dans un second temps, seront plus exigeants. Cela passe également par l'élaboration d'une stratégie numérique responsable dans les territoires, qui fait l'objet d'un nouveau chapitre. Je me réjouis de l'adoption de l'amendement que nous avions déposé en commission visant à prendre en compte l'empreinte environnementale du numérique au sein des plans N'oublions pas toutefois les responsabilités du secteur économique. Les mesures de cette proposition de loi semblent donc aller dans le bon sens s'agissant des nouvelles obligations en matière d'écoconception des sites web les plus fréquentés, de la création d'un référentiel général de l'écoconception, de l'avantage fiscal prévu pour les centres de données moins énergivores ou encore des nouveaux engagements de réduction des impacts environnementaux des réseaux. La préservation de l'environnement doit être prise en compte par tous les acteurs de la filière et la régulation de l'Arcep, en la matière, doit se faire avec davantage de contraintes.

signe aussi d'un dialogue que je crois constructif avec le Gouvernement, qui semble avoir pris le sujet en main et verra, je l'espère, cette initiative parlementaire comme une opportunité à saisir. C'est en tout cas la position du groupe RDSE, qui salue ce travail équilibré et souhaite voir émerger au plus vite une véritable politique publique de sobriété du numérique, sans pour autant freiner les progrès économiques, sociaux et écologiques incontestables qu'il engendre. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas. Madame la présidente,

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la démarche qui a présidé à la création de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique et à la rédaction de cette proposition de loi semble pertinente. Nous saluons le travail réalisé par le président et le rapporteur de la mission, tout comme celui de la commission sur le sujet. Cette proposition de loi s'articule pleinement avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, mais aussi avec la feuille de route du Gouvernement, largement convergente avec le contenu de ce texte. Notons également l'adoption au niveau européen d'une proposition de résolution à ce sujet en novembre dernier. Cette prise de conscience est celle de l'urgence écologique qui nous oblige collectivement à tracer les contours d'une société plus économe en ressources et plus sobre en consommation énergétique. La France, qui s'est engagée à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à arriver à la neutralité carbone en 2050, doit prendre des mesures fortes. À ce titre, le secteur numérique semble un levier puissant de transformation : si le numérique constitue aujourd'hui seulement 2 % du total des émissions en 2019 dans notre pays, cette empreinte pourrait augmenter de 60 % d'ici à 2040 si rien n'est fait. Pour autant, les dispositions contenues dans cette proposition de loi, après l'examen du texte en commission, semblent en retrait par rapport aux objectifs affichés. de loi risque malheureusement d'être peu opérante face à la complexité des enjeux industriels et stratégiques, notamment en matière de souveraineté numérique, mais également face au niveau d'action nécessaire lié à l'immatérialité de cette économie et à la globalisation des échanges. échanges. Comme l'exposé des motifs le souligne, les impacts carbones du numérique sont liés essentiellement à la production des terminaux, production principalement localisée en Asie. Relocalisation de l'économie, développement d'une filière industrielle au niveau européen, changement des règles du libre-échange, abrogation des accords commerciaux fondés sur le social, économique et environnemental, autant de sujets qui sont alors incontournables pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique et qui ne sont pourtant pas évoqués dans cette proposition de loi. Il en est de même de la nécessaire réflexion à l'échelle internationale sur l'accès à la ressource en eau et sur la gestion des terres rares dont sont particulièrement friands ces appareils Faute de s'attaquer au modèle économique libéral de production et de proposer des alternatives permettant de garantir tout au long du processus de production et d'utilisation des équipements électroniques numériques un usage plus vertueux, les dispositions contenues dans cette proposition de loi risquent de perdre en opérationnalité.

il y a un peu plus d'un an lors de l'examen de la loi sur l'économie circulaire. Ce texte a marqué de nombreuses avancées, y compris grâce à l'adoption d'amendements émanant de notre groupe. Il en est ainsi de la lutte contre l'obsolescence logicielle. Nous sommes à ce titre surpris d'un changement de pied de la majorité sénatoriale sur certains sujets comme l'extension de la garantie légale ou la révision du taux de TVA. Nous proposerons d'aller plus loin et formulerons des propositions qui, à l'époque, n'avaient pas trouvé de majorité. Nous espérons qu'elles trouveront aujourd'hui une issue plus favorable. Concernant les obligations formulées auprès des entreprises, nous ne pouvons que nous ne pouvons que constater que la portée des dispositions initialement proposées a été largement revue à la baisse, notamment au travers la suppression des articles 17 à 20.

contourner de manière habile le caractère contraignant de ces mesures au bénéfice d'un référentiel à la portée plus souple et à la valeur juridique floue. Ses modalités d'élaboration sont finalement renvoyées aux ingénieurs alors que ces questions sont avant tout politiques.

Pour finir et élargir le débat, et alors que l'impact environnemental de ces usages numériques est très lié aux Gafam, pourquoi ne pas revenir ici sur leur imposition afin qu'ils contribuent réellement aux politiques publiques contre le changement climatique ? Il nous semble prioritaire de sortir de l'impunité ces grandes multinationales qui n'ont, en l'état, aucune raison de s'orienter vers la sobriété numérique et qui ne contribuent pas à l'effort collectif pour la transition écologique. Malheureusement, nous doutons que cette proposition de loi change la donne en la matière

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, de nombreux spécialistes, de nombreux industriels, de nombreuses associations environnementales sont d'accord pour dire que le numérique constitue un atout idéal pour résoudre en partie la problématique climatique. La proposition de loi que nous étudions ce jour prouve que le numérique occupe une place importante dans les transitions écologique et énergétique. Comme cela a été souligné, le numérique pourrait représenter à l'horizon de 2040 près de 7 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. Nous saluons le travail parlementaire effectué lors de la mission d'information, qui a rendu ses conclusions en juin dernier. La traduction législative que nous étudions a déjà été améliorée lors de l'examen par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Cette proposition arrive à un moment opportun, c'est maintenant que nous devons nous emparer de ce sujet. Il est devenu évident, au vu de l'implication de chacun dans le numérique et ses usages, que tous y participent : les consommateurs, les entreprises ou encore le secteur public. Ainsi, nous prenons collectivement conscience de l'impact du numérique dans nos usages quotidiens et nos choix de consommation. À ce titre, la création d'un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique sera utile pour anticiper les évolutions futures et les contraintes auxquelles nous devrons faire face. La durée de vie et la réutilisation des terminaux que nous utilisons pour avoir accès au numérique sont un des enjeux majeurs. À juste titre, la commission est revenue sur le renversement de la charge de la preuve prévu à l'article 6 du texte relatif à l'obsolescence programmée. La nouvelle rédaction de l'article, qui vise à supprimer l'un des critères d'intentionnalité constituant le délit d'obsolescence programmée, est une réelle transformation du mécanisme. Autre point qui a retenu notre attention et qui a fait l'objet d'un travail important en commission : l'écoconception des sites web. Le cadre général proposé regrouperait plusieurs critères dont nombre d'entre eux semblent nécessaires. J'entends par là particulièrement ce qui a trait à l'affichage et aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs. Les vidéos qui se déclenchent automatiquement à l'ouverture d'un réseau ou d'une page web, en plus d'être consommatrices de données et d'énergie, nuisent bien souvent à la navigation des utilisateurs. Enfin, je terminerai mon propos en saluant la volonté des auteurs de ce texte de réduire les impacts environnementaux des centres de stockage des données numériques. Ces centres seront de plus en plus nécessaires : nous devons donc réduire leur empreinte au maximum. Cette proposition de loi, exemple très parlant du travail d'avant-garde que peut produire le Sénat, et l'examen que nous allons en faire marquent l'importance de la réflexion et de l'action que nous menons dans cette chambre, au bénéfice des territoires. Je forme le voeu qu'elle constitue une base solide à notre stratégie nationale vers un numérique responsable qui pourra en inspirer d'autres. La parole

d'État, mes chers collègues, les enjeux liés à l'empreinte environnementale du numérique ont longtemps été minimisés, voire ignorés. Alors que, jusqu'ici, on était surtout sensibles aux gains de productivité résultant du numérique, à ses effets de substitution, pour reprendre l'expression de M. le secrétaire d'État, on prend à présent conscience de sa contribution en forte croissance au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources abiotiques, à des tensions sur l'eau douce et à diverses formes d'agressions des écosystèmes. Selon tous ces critères, en 2019, l'impact planétaire du numérique représentait deux à trois fois l'empreinte environnementale tous secteurs confondus de la France, et ce n'est pas fini Entre 2010 et 2025, la taille de l'univers numérique va au moins tripler et ses impacts environnementaux vont au moins doubler. « Au rythme actuel, le numérique sera considéré comme une ressource critique non renouvelable en voie d'épuisement d'ici moins d'une génération », selon l'expert indépendant Frédéric Bordage. Malgré les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris, il n'existe à ce jour aucune législation qui permette de contrôler, de réguler ou de réduire les impacts environnementaux du numérique. C'est un vide juridique criant. Face à ce vide, la mission d'information sénatoriale et cette proposition de loi qui en a découlé sont particulièrement opportunes. Le groupe écologiste salue ce texte, qui témoigne d'un travail transpartisan pour le moins riche et ambitieux. Il est en phase avec des propositions portées par le Conseil national du numérique et par la Convention citoyenne pour le climat. Il s'inscrit dans le sillage de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Ce n'est Ce n'est hélas ! pas le chemin que semble prendre le récent projet de loi climat du Gouvernement, qui ne comble pas ce manque de régulation environnementale du numérique. Certes, le Gouvernement a présenté une feuille de route, mais sa mise en oeuvre concrète n'est pas claire. La présente proposition de loi est donc, je le répète, particulièrement opportune. Il s'agit d'engager une transition du numérique par des modes de production, de commercialisation et de consommation qui privilégient la sobriété, un usage raisonné et plus respectueux de l'environnement. Cette transition du numérique, c'est ce que souhaitent les écologistes. Monsieur le secrétaire d'État, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure qui vous visiez en parlant dans ce débat de postures idéologiques réactionnaires et en évoquant- j'en ai été étonné -un slogan pétainiste. Carrément ! Sachez que le groupe écologiste ne se reconnaît absolument pas Revenons-en au fond. Ce texte novateur a de nombreux points forts. Il vise particulièrement les producteurs et les fournisseurs en augmentant leurs obligations en matière de reconditionnement, de recyclage, de réparation et de conformité. À ce titre, la lutte contre l'obsolescence programmée et l'augmentation de la durée légale de conformité de deux à cinq ans seraient des avancées majeures, en particulier dans le contexte de déploiement de la 5G, qui remet en question la viabilité des équipements numériques actuels. Il permettrait d'apporter plus de transparence sur les stratégies des entreprises et consacrerait l'écoconditionnalité, ainsi que des engagements pluriannuels contraignants. Le groupe écologiste proposera de renforcer ce texte D'abord, il est essentiel que les objectifs visés soient clairs : il s'agit donc d'obtenir l'inscription d'objectifs propres au numérique dans la stratégie nationale bas-carbone, la SNBC. Cette dernière doit prévoir un volet spécifique à ce secteur et définir un budget carbone fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous proposons aussi l'évaluation de l'impact environnemental de la 5G par l'observatoire créé par la présente loi : le rapport remis juste avant Noël par le Haut Conseil pour le climat montre clairement cette nécessité. Nous mettons également au débat, par voie d'amendements, la question du gâchis de consommation d'énergie des dispositifs publicitaires numériques. Nous demandons de rétablir l'article 19 dans sa rédaction initiale afin de mettre fin au lancement automatique des vidéos lors de la consultation de sites internet, sauf dérogation. Nous regrettions la suppression en commission de l'obligation pour les opérateurs téléphoniques de moduler les forfaits proposant des données internet afin d'encourager une consommation raisonnée le wifi ou le filaire. Nous souhaitons donc renforcer l'article 15 pour enrayer la croissance des consommations réseaux à laquelle nous expose le déploiement de la 5G. Enfin, pour lutter contre l'obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des terminaux, nous proposons de travailler le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques, voire d'expérimenter dans des territoires volontaires un dispositif de consigne. Ces propositions sont fidèles à l'esprit du texte, appuient ses dispositions et, vous l'avez compris, ne visent qu'à le consolider et à assurer son efficacité. L'enjeu, aujourd'hui, est d'adopter un usage raisonné du numérique et de préserver nos ressources pour garantir un avenir viable.

Le numérique, nous le disons depuis maintenant un certain nombre d'années dans cette assemblée, est indispensable à nos concitoyens, à l'attractivité de nos territoires, au développement économique et à l'innovation. Ses atouts ne doivent pas pour autant nous faire mettre de côté son impact environnemental, incontestablement insuffisamment pris en compte jusqu'à présent. Les usages numériques ne sont pas sans conséquence sur l'environnement en termes d'émission de gaz à effet de serre, de consommation énergétique ou d'utilisation des ressources. Ce constat longtemps occulté a conduit la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat à mettre en place à la fin de 2019 une mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique. Ses travaux ont abouti à un rapport de grande qualité. Je salue particulièrement le travail de Patrick Chaize, de Jean-Michel Houllegatte et de Guillaume Chevrollier. Ce rapport a notamment permis pour la première fois une évaluation de l'empreinte carbone numérique dans notre pays.

Il souligne donc la nécessité de mettre en place une politique de sobriété numérique pour concilier transition numérique et transition écologique, toutes deux indispensables. C'est le sens de la feuille de route déclinée par le rapport, qui prévoit vingt-cinq mesures, reprises- pour celles qui relèvent du niveau législatif -dans cette proposition de loi. Le présent texte, dont j'ai l'honneur d'être coauteur et qui a été amélioré par la commission au fond et celle saisie pour avis ainsi que par le travail des rapporteurs, prévoit que notre pays se dote d'outils pour anticiper l'impact du numérique sur le climat et rendre son développement compatible avec nos engagements internationaux.

Ainsi, dans le prolongement de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ainsi que des apports de notre assemblée sur ce texte, la présente proposition de loi renforce les outils de lutte contre l'obsolescence programmée, privilégie les produits durables dans la commande publique, améliore la collecte des produits numériques et favorise le développement du marché de seconde main. main. Elle prévoit également d'inciter aux usages numériques vertueux, en imposant un référentiel général de l'écoconception aux sites internet qui génèrent le plus de trafic. Elle aborde enfin la question préoccupante de l'impact environnemental des réseaux en dotant notre pays de moyens d'anticiper et de réguler cet impact, qui devrait augmenter avec les réseaux de nouvelle génération. À cet égard, je rappellerai que, conscient des enjeux environnementaux de la 5G, le président du Sénat a saisi à notre demande le Haut Conseil pour le climat (HCC) afin qu'une estimation de son impact soit réalisée. Le rapport du HCC est plutôt alarmant puisqu'il estime que cette génération de réseau entraînera une « augmentation significative » de l'empreinte carbone du numérique. Il est donc regrettable que le Gouvernement n'ait pas, comme nous le demandions, effectué une évaluation préalable au déploiement de la 5G. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, nous devons faire en sorte que l'indispensable développement du numérique s'effectue de manière sobre, responsable et respectueuse de l'environnement. C'est un enjeu essentiel qu'il nous appartient, ensemble, de relever. Tel est l'objectif de cette proposition de loi. La parole

l'initiative prise par nos collègues Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte permet d'apporter un éclairage novateur, judicieux et pertinent sur l'empreinte environnementale du numérique. Qu'ils en soient remerciés Ce sujet appelait depuis longtemps un débat et un travail de fond, dont la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est opportunément saisie. Le soutien de 130 cosignataires en confirme l'importance. Toutes les politiques publiques devraient désormais s'inscrire dans une démarche d'évaluation environnementale afin de conditionner leur mise en oeuvre. Cela semble s'imposer pour le numérique, qui prend une dimension particulière avec la montée en puissance de la 5G, avec comme corollaire une évolution significative des usages, des moyens et des outils. L'évolution d'une prise de conscience générale s'est traduite dans plusieurs rapports et propositions. Je citerai climat et du Haut Conseil pour le climat, sur l'empreinte environnementale de la 5G, de l'Arcep, pour des politiques numériques plus soutenables. Aussi cette proposition de loi contribue-t-elle à ouvrir objectivement un débat trop souvent marqué par des radicalités peu éclairantes, souvent réductrices, qui ne permettent pas d'envisager ces problématiques dans toute leur complexité, et cela notamment du fait de l'absence de données environnementales, d'outils pour les collecter et d'évaluations. Comment faire de la transformation numérique un accélérateur positif de la transition écologique, si ce n'est en accompagnant et en progressant collectivement, pour conforter les démarches d'évaluation environnementale ? L'évaluation est consubstantielle des politiques de développement durable. Reconnaissons dans ce domaine nos faiblesses, nos carences et la nécessité d'établir de nouveaux référentiels communs pour s'appuyer sur des indicateurs partagés, pour mieux mesurer les impacts et agir en conséquence sur les usages, notamment par une meilleure information et une responsabilisation des acteurs et des usagers. mieux réguler en s'appuyant sur des données objectives en créant, à l'article 3 du texte, un observatoire des impacts environnementaux du numérique, mais également sur les plus-values et gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique. Une approche globale est proposée dans ce texte. Elle doit fournir un cadre vertueux en intervenant sur l'ensemble de la chaîne numérique- des équipements aux logiciels, jusqu'aux centres de données -et en abordant les questions de durabilité, de réemploi et d'obsolescence, souvent dénoncée et pourtant si mal régulée. L'équilibre des propositions se fait par des mesures d'incitation pour susciter la prise de conscience et des mesures contraignantes afin d'imposer aux opérateurs de réduire réellement leur impact environnemental. L'approche normative est confortée notamment, quant à l'obsolescence, dans une logique de responsabilité sociétale des acteurs plutôt qu'au travers d'un cadre exclusivement contraignant. Enfin, le texte approfondit la responsabilité sociétale de tous les acteurs : particuliers, entreprises, collectivités et territoires. La responsabilité sociétale des entreprises doit en effet étudier les conditions de son extension à la sobriété numérique et il est essentiel que tous les acteurs du secteur public, comme du secteur privé, s'inscrivent dans ces orientations pour une évolution favorable du sujet. Les territoires sont évidemment le maillon indispensable d'une politique d'équilibre pour une couverture numérique ambitieuse et le respect de l'environnement, une convergence entre transition numérique et transition écologique. Les amendements socialistes adoptés en commission se sont traduits dans un nouveau chapitre intitulé « Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires », en affirmant une gouvernance territoriale : en permettant aux collectivités de plus de 50 000 habitants d'inscrire une stratégie numérique dans leur rapport de redevabilité sur le développement durable ; en intégrant les dans les systèmes énergétiques locaux et dans les plans climat-air-énergie territoriaux en mobilisant l'achat public pour réduire l'empreinte carbone du numérique au sein des schémas de promotion des achats publics responsables. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez invoqué dans un premier temps l'urgence du déploiement de la 5G afin d'éviter une perte de compétitivité et d'attractivité pour notre pays. Dans un second temps, vous avez défendu l'utilité des nouvelles technologies numériques pour accélérer la transition écologique. Notre difficulté, nous le savons, réside dans ce que les modèles de leur développement s'appuient sur les usagers ainsi que sur la multiplication et la diversité de l'offre en vue de trouver une rentabilité. Ces enjeux économiques et financiers ne doivent pourtant pas nous détourner de nos objectifs environnementaux, aujourd'hui essentiels. L'enjeu primordial de ce texte est de valoriser le numérique en maîtrisant son empreinte environnementale pour qu'il soit un outil de progrès, atout d'une transition écologique et non pas obstacle aux enjeux climatiques. L'initiative du Sénat sur le sujet, qui a été très suivie, marque la nécessité de répondre rapidement au défi d'une politique numérique responsable sur le plan environnemental. Cette proposition de loi apporte les premières solutions pour envisager une meilleure régulation, en informant et en responsabilisant tous les acteurs, opérateurs et citoyens, et en introduisant une approche territoriale indispensable.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer Patrick Chaize, auteur de la proposition de loi, et les rapporteurs pour avis et au fond, Anne-Catherine Loisier, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, pour le travail accompli et la pédagogie dont ils ont réussi à faire preuve pour expliquer cette problématique « contre-intuitive ». En effet, contrairement à ce que certains usagers imaginent- cela a été rappelé par nos rapporteurs -, le numérique n'est pas immatériel. Il laisse une empreinte sur l'environnement et celle-ci est malheureusement exponentielle : 2 % des émissions de gaz à effets de serre aujourd'hui en France, et 7 % dans vingt ans. Faire émerger des pratiques plus vertueuses chez les acteurs du numérique et chez les consommateurs s'impose pour réguler notre empreinte, sans toutefois fragiliser les filières. C'est là toute l'agilité de nos collègues équilibristes qui sont parvenus à formuler des propositions de maîtrise des impacts environnementaux sans handicaper nos entreprises nationales. Les priorités de ce texte sont claires et intelligibles : informer, éduquer, lutter contre le renouvellement des terminaux, promouvoir des usages écologiquement vertueux et développer des centres de données moins énergivores. Parce que ces nouvelles pratiques s'imposent à tous, aux acteurs du numérique comme aux citoyens, nous ne pouvons nous contenter d'ordonnances techniques de transposition des directives européennes. La représentation nationale doit en débattre. Plusieurs points ont en particulier retenu mon attention. Il s'agit tout d'abord de la mise en oeuvre de l'article 16, qui rend obligatoire l'écoconception des sites web et des services en ligne publics, mais aussi de certaines entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par décret en Conseil d'État. Je regrette cette restriction qui écarte certaines entreprises. L'écoconception des environnements web ne doit pas être perçue comme un surcoût de conception. Développer « écoconçu » revient à appliquer une méthodologie précise et rigoureuse qui ne demande ni plus de temps ni plus d'argent. Une directive à l'endroit de toutes les entreprises me semble donc souhaitable pour assurer la sobriété numérique, raison pour laquelle je proposerai un amendement en ce sens. Toujours Toujours à l'article 16, nos rapporteurs ont souhaité reporter à 2023 l'entrée en vigueur du dispositif. Ce report ne me semble pas souhaitable dans la mesure où il existe d'ores et déjà beaucoup de matière- rapports, recommandations, etc. -pour établir le référentiel d'écoconception d'un site web. La formation des différents acteurs de l'écoconception et les démarches d'amélioration sont en ordre de bataille, et elles doivent se poursuivre. Il semble donc inutile, voire regrettable, de faire attendre un marché qui s'est déjà structuré et qui a développé des solutions. Reporter les efforts à une échéance lointaine pénaliserait finalement davantage les acteurs qui se disent aujourd'hui « prêts ». C'est pourquoi je défendrai également un amendement visant à supprimer ce délai. Pour terminer sur l'obligation d'écoconception des sites, ne serait-il pas également souhaitable d'y associer des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ? Cet ajout ne rallongerait en aucun cas la conception des sites web et il permettrait une portée RSE globale. Sur le volet relatif aux centres de données, je proposerai également un amendement visant à faire bénéficier du tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) les acquéreurs de à climatisation adiabatique qui permettent des économies d'énergie substantielles. C'est aussi un enjeu de développement économique important pour nos territoires, auxquels le Sénat porte toujours une attention particulière. Avec cette proposition de loi, le Sénat fait véritablement oeuvre utile. Il propose des solutions adaptées et concrètes au défi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.

la relation entre numérique et environnement est ambivalente. D'un côté, la numérisation est présentée comme un outil incontournable de lutte contre le réchauffement climatique. En effet, l'intelligence artificielle et le sont aujourd'hui mobilisés pour mener la transition énergétique. Compteurs et réseaux intelligents vont avoir la capacité d'ajuster en temps réel l'offre à la demande d'électricité et, ainsi, d'offrir le pilotage nécessaire au déploiement d'énergies d'énergies renouvelables par nature intermittentes, comme l'éolien ou le solaire. Le numérique sera la clé d'amélioration de l'efficacité énergétique de toute l'économie. Mais, d'un autre côté, il faut bien reconnaître que les vertus environnementales du numérique ne sont encore qu'en puissance. Car la numérisation est de plus en plus énergivore. L'ensemble des équipements permettant de traiter, de stocker et d'échanger des données absorberait déjà entre le quart et la moitié de l'électricité mondiale, générant entre 2 % et 10 % des émissions mondiales de CO2.

Le numérique ne pourra donc tenir ses promesses écologiques que si l'on s'emploie à le décarboner en amont. C'est bien pourquoi le présent texte n'a rien d'anodin. Nous tenons à souligner son caractère précurseur. D'ailleurs, le Haut Conseil pour le climat en a indirectement validé les conclusions dans son avis du 19 décembre sur la 5G. Au passage, c'était la première fois que le HCC était saisi par une assemblée parlementaire. C'est aussi la première fois que le législateur se saisit en France de ce sujet d'avenir, d'autant plus déterminant que la problématique entre en résonnance avec celle de l'autonomie et de la souveraineté numérique de notre pays. Les conclusions de la mission d'information ayant conduit à la présente proposition de loi sont claires : plus de 80 % des impacts environnementaux du numérique en France sont dus aux terminaux numériques. Et pourquoi les terminaux numériques ont-ils un tel impact ? Parce qu'ils ne sont pas fabriqués en France ! Importer nos terminaux, c'est à la fois importer de la dépendance économique et de la pollution. Le texte aborde de front le problème dans ses articles 6 à 14, qui nous semblent constituer son apport principal. La dimension pédagogique du sujet a certes son importance à long terme. Mais aujourd'hui, c'est la limitation de l'importation et du renouvellement des terminaux qui constitue le nerf de la guerre. Pour conclure, je dirai un mot de l'énorme travail effectué en commission pour compléter la première mouture du texte. Nous ne pouvons que saluer les avancées réalisées pour renforcer la lutte contre l'obsolescence programmée, promouvoir l'écoconception des sites web ou renforcer la sécurité juridique du texte. Mais, dans cet hémicycle, une dimension nous tient plus que tout à coeur : la dimension territoriale. On ne rendra pas le numérique durable sans stratégies numériques responsables sur les territoires. Grâce à la décentralisation, le numérique est devenu le phénomène central du désenclavement de la ruralité profonde. On ne le verdira aussi que grâce à la décentralisation. C'est bien ce que prévoit maintenant le texte en donnant mission aux agglomérations, aux départements et aux régions de décliner à leur échelle la feuille de route du verdissement du numérique. Vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte. Monsieur le secrétaire d'État, nous espérons vraiment que, à la faveur de son examen, le Gouvernement s'emparera de ce sujet. La présente proposition de loi devra être complétée, car elle n'aborde la durabilité du numérique que sous l'angle des émissions de CO2. Or l'empreinte environnementale du numérique pèse aussi par sa consommation de matières premières, en particulier de métaux et de terres rares.

cette proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique pose pour la première fois ce débat au niveau législatif et opte pour une régulation renforcée. Je tiens à saluer préalablement le travail mené sur le long terme, avec l'ensemble des groupes politiques, et conclu par le rapport nos collègues. Nos concitoyens connaissent les nombreux avantages qu'apporte le numérique dans leur quotidien : facilité des échanges, des communications instantanées et un meilleur partage de l'information. Mais ont-ils conscience des impacts sur notre vie et l'environnement liés à la fabrication et l'utilisation de nos outils numériques ? Notons une multiplication des équipements, des équipements, une consommation d'énergie qui représente 4 % du total de l'énergie consommée mondialement. Cette prise de conscience collective est nécessaire pour réfléchir sur nos usages, plus particulièrement au niveau de l'État et de nos collectivités territoriales. Cette proposition de loi doit être une première pierre, nous devons montrer l'exemple. Il ne suffit pas de modifier la loi, nous devons modifier nos comportements, nos habitudes.

de loi fixe un premier cadre : à nous de le développer partout, en commençant par nos entreprises. Une évolution du champ de la RSE, avec un caractère plus incitatif, serait souhaitable. En effet, malgré un indéniable effet pédagogique, les obligations issues des travaux sur la RSE restent limitées dans les entreprises. L'article 4 prévoit d'inscrire l'impact environnemental du numérique dans le bilan RSE des entreprises. Cette mesure, complétée par

les entreprises de plus de 500 salariés et les collectivités locales ou leurs groupements de plus de 50 000 habitants. Mes chers collègues, la loi du 10 février 2020 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire porte des dispositions incitatives en faveur de biens plus durables. Nous allons donc dans le bon sens, avec la mise en place d'un indice de réparabilité sur les équipements et, à compter de 2024, d'un indice de durabilité. Au coeur de cette économie circulaire, et afin de faciliter le recyclage et de prolonger la durée de vie des équipements- sachant que la prolongation de l'utilisation d'un ordinateur de deux à quatre ans améliore son bilan environnemental de 50 l'article 6 tend à rendre le dispositif qui définit et sanctionne l'obsolescence programmée plus dissuasif, en inversant la « charge de la preuve ». Il incomberait au producteur, et non plus au consommateur, de prouver que la réduction de la durée de vie du terminal n'est pas délibérée et qu'elle découle d'éléments objectifs étrangers à toute stratégie d'augmentation du taux de remplacement. C'est un article très important puisque, aujourd'hui, très peu de poursuites au titre de l'obsolescence programmée ont pu être réellement engagées et donner lieu à des sanctions. Alors que 10 milliards de téléphones portables ont été vendus depuis 2007, l'article 7 intègre l'obsolescence logicielle dans la définition donnée à l'obsolescence programmée. C'est une avancée. Faisons en sorte que la transition numérique ne laisse pas certains de nos concitoyens au bord de la route. Profitons de l'avancée de cette transition pour accompagner les usagers

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la mission d'information conduite par nos collègues Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, relative à l'empreinte environnementale du numérique en France, a identifié un véritable angle mort de notre politique de lutte contre le réchauffement climatique. Or, si nous voulons atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris, nous devons nous pencher sur la pollution du secteur numérique. En ce sens et à partir des vingt-cinq propositions figurant dans le rapport de nos collègues, nous avons été nombreux à cosigner cette proposition de loi. Le caractère transpartisan de ce texte, le rôle majeur du Sénat comme défricheur d'un champ émergent encore mal appréhendé, la dimension anticipatrice et préventive de cette proposition de loi lui confèrent un caractère novateur à divers titres.

Pour autant, d'autres dimensions introduites par cette proposition de loi me semblent emblématiques de l'évolution nécessaire de nos politiques publiques et de notre responsabilité collective autour de l'information, de la formation et de la prévention. l'information et la formation, tout d'abord, il s'agit d'assurer un retour à la confiance dans la parole du politique, au sein d'une société chaque jour davantage frappée par des informations erronées et non hiérarchisées provenant de sources invérifiables, et où les ont envahi notre espace. À ce titre, l'éducation des plus jeunes dès l'école à une utilisation responsable des outils numériques constitue en soi un projet de société. De même, la conditionnalité introduite dans le parcours diplômant des ingénieurs en informatique à une certification en écoconception logicielle me semble être un élément essentiel. La prévention, ensuite, constitue une innovation majeure pour nos politiques publiques. La plupart du temps, nous agissons en réaction, en correction. Là, nous avons la possibilité avec cette loi d'anticiper, de prévenir.

Nous le savons. Nous pouvons donc agir sur les divers leviers proposés : éducation, limitation du renouvellement du matériel, développement des usages écologiquement vertueux. Alors, n'hésitons pas ! Notre responsabilité collective est bien là. J'en viens donc à la responsabilité des entreprises en matière de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Il me semble que nous pourrions aller plus loin encore. La prise de conscience par les entreprises de cette nouvelle dimension environnementale tendant à mieux informer, mieux valoriser les actions engagées, mieux reconnaître leur responsabilité sociale et environnementale, est déjà bien engagée. Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), qui ambitionnait de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois, a fait l'objet d'une loi promulguée le 22 mai 2019. L'entreprise participe historiquement à l'intérêt général, étant moteur du progrès économique et technologique, créateur de lien social et lieu d'accomplissement personnel. Comment l'État peut-il jouer un rôle dans cette refondation de l'entreprise et de ses missions ? Nous avons déjà commencé à y répondre ; il nous faut aller plus loin. La France fait en effet déjà figure de pionnier sur ces sujets.

Afin d'accélérer cette dynamique, la loi Pacte a acté dans le droit le fait que l'entreprise a un deuxième objectif, parallèlement à sa profitabilité : sa raison d'être. Celle-ci peut se définir par l'expression d'un futur désirable pour le collectif. Cette raison d'être peut notamment permettre de renforcer l'engagement des salariés, en étant porteuse de sens. Ainsi, la loi Pacte a arrimé l'entreprise dans le XXI siècle en consacrant sa responsabilité sociétale, qui sera désormais décryptée à travers trois niveaux d'engagement : la considération des impacts sociaux et environnementaux liés à son activité la réflexion sur son environnement à long terme ; enfin, le statut de « société à mission ». On entend ici par « mission » une « raison d'être » à plus-value sociétale que se donne l'entreprise. Plus concrètement encore, il peut s'agir d'inventer de nouveaux modèles de consommation plus responsables, ou encore de contribuer à la reforestation d'un pays fournisseur, ou justement de réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est essentiel, la consommation électrique du numérique

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer les travaux de la mission d'information sur l'empreinte carbone du numérique, laquelle était jusqu'ici sous-évaluée et quasiment absente des objectifs fixés dans les accords sur le climat. Cette évaluation sur toute la chaîne de production et de consommation du numérique permet de proposer, en toute connaissance de cause, des solutions concrètes et des alternatives à la surconsommation de ces produits. En adoptant une démarche pragmatique, cette proposition de loi répond à la nécessité de rendre visibles les impacts cachés de ce secteur dématérialisé. En amont, la majeure partie de ces impacts proviennent de la fabrication des équipements, qui est délocalisée. De même, les réseaux mobiles et les data centers, dont l'empreinte carbone est très élevée, demeurent invisibles pour l'utilisateur final. Enfin, contrairement aux idées répandues, la multiplication des usages entraîne une surconsommation d'énergie, qui annule les gains générés dans les premières années. L'information du public et la prise de conscience des consommateurs sont donc indispensables, mais pour autant insuffisantes. Le temps des injonctions culpabilisantes étant révolu, ce texte montre la bonne voie en proposant des solutions et des outils incitatifs auxquels les consommateurs peuvent choisir d'adhérer. En nous appuyant, à la fois, sur l'innovation et sur la réglementation, nous avons les moyens de réguler l'obsolescence programmée des appareils et des logiciels, de rallonger la durée des usages ou encore d'inciter à l'achat de produits reconditionnés et moins énergivores. En effet, depuis le 1 janvier 2021, les vendeurs de smartphones et d'ordinateurs sont obligés d'afficher un indice de réparabilité sur ces équipements, selon l'article 16 de la loi sur l'économie circulaire, en indiquant clairement sur quelles données reposent leurs calculs. Par ailleurs, cette loi a inscrit dans le code de l'environnement l'interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil. Autrement dit, il sera désormais illégal de programmer la fin de vie d'un produit et d'empêcher sa réparation par quelque moyen que ce soit. La proposition de loi du Sénat s'inscrit dans la même logique d'efficacité avec des mesures qui reposent à la fois sur des gains écologiques et économiques. En étant complémentaires, ces deux piliers peuvent réellement inciter chaque acteur à modifier ses pratiques, qu'il s'agisse des particuliers, des entreprises ou des collectivités. Enfin, la réparation de ces produits est créatrice d'emplois non délocalisables. Dans le Bas-Rhin, par exemple, les collectes d'anciens téléphones portables ou de chargeurs sont organisées

ces filières représentent un enjeu de taille dans la crise actuelle. Les articles 12 à 14 du texte y sont consacrés, notamment par la création d'un taux de TVA à 5,5 % pour les produits reconditionnés. Aujourd'hui, ce potentiel est encore loin d'être très utilisé selon l'étude réalisée par OpinionWay en juillet 2019 pour l'Alliance française des industries du numérique : seulement 4 à 8 millions d'appareils usagés sont reconditionnés chaque année. En revanche, une centaine de millions d'appareils qui pourraient être réparés dorment dans les tiroirs des Français. Le secteur numérique n'a pas qu'une empreinte environnementale, il a aussi une empreinte sociétale, les deux étant liées. En conclusion, nous avons avec ce texte une feuille de route claire et précise qui permet d'impliquer les consommateurs, d'une part, et d'engager la responsabilité des producteurs, d'autre part. Pour ces différentes raisons, je voterai cette proposition de loi. La

Cinq ans ont passé depuis l'Accord de Paris et l'engagement historique que nous avions pris en faveur du climat : il est plus que temps d'accélérer ! Je rappelle à quel point le Sénat est fort lorsqu'il unit ses forces. Ce texte est un texte transpartisan

Ce texte est aussi très important dans la perspective de nos futurs débats sur le texte relatif au climat. À ce stade, l'avant-projet de loi ne comprend pas de mesures sur la question de l'empreinte environnementale du numérique il pourra ainsi être considérablement enrichi par l'adoption de cette proposition de loi. Ce texte répond également à une très forte attente de nos concitoyens, lesquels veulent avoir accès à un numérique vertueux, qui est un outil puissant au service de la transition écologique. Je souhaiterais souligner le travail important et exigeant qui a été réalisé par notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur cette proposition de loi. Il y eut, d'abord, une mission d'information, dont je salue les anciens membres, comme Hervé Maurey, les rapporteurs, Jean-Michel Houllegatte et Guillaume Chevrollier, et bien entendu le président Patrick Chaize. Le texte a été examiné en commission, avec l'éclairage important de la commission des affaires économiques, saisie pour avis, dont je salue la rapporteure, Anne-Catherine Loisier, Loisier, et largement enrichi. Je me réjouis de constater que personne n'a aujourd'hui souhaité revenir sur les principales orientations retenues, ce qui montre que la philosophie du texte fait l'objet d'un fort consensus.

Rudy Reichstadt, membre de l'Observatoire des radicalités politiques et fondateur du site Conspiracy Watch, évoquait récemment la rencontre entre une offre idéologique complotiste mondialisée et des capacités matérielles historiques, rendant possible sa propagation. Au travers de ce qu'on appellera très imprécisément « les écrans », cette mal-information, cette surconsommation d'informations que nous pourrions comparer à de la malbouffe, a un coût cognitif, sanitaire et environnemental.

Membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, il défend la piste éducative et l'apprentissage de l'esprit critique pour faire face à un marché totalement dérégulé. Reprendre notre souveraineté écologique et cognitive passera donc par une éducation ciblée et des mesures fortes préventives- nous en débattrons à l'article 16. Dans le cadre de l'obligation d'écoconception des services numériques, le décret pris en Conseil d'État devra prendre en compte cet impératif de protection de notre attention, notamment dans le cadre du référentiel général qui sera mis en oeuvre. En conclusion, et c'est le sens de mon intervention, je pense qu'une attention préservée, mieux armée et mieux prévenue sera un levier indispensable à une consommation plus

qui peut paraître symbolique, mais qui a en réalité une grande importance. Si le numérique a permis de maintenir l'éducation et la formation de la jeunesse pendant la crise sanitaire, l'explosion de son utilisation n'est pas sans poser problème- c'est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Tablettes, ordinateurs, smartphones, serveurs sont fabriqués à partir de métaux, dont l'extraction, faite dans des pays peu respectueux des normes environnementales et sociales, à un rythme qui mène à un épuisement de ces ressources, est extrêmement polluante. Par ailleurs, l'énergie nécessaire à leur chaîne de production est majoritairement fossile. Le numérique, c'est aussi une consommation électrique qui explose, avec 6 à 10 % de la consommation électrique mondiale. Enfin, lorsqu'ils ne fonctionnent plus ou sont devenus obsolètes, les objets numériques deviennent des déchets très polluants et peu valorisés. Tout cela s'apprend, et il est impératif que les jeunes aient conscience de l'ensemble de ces impacts environnementaux. C'est pourquoi l'école a un rôle majeur à jouer pour sensibiliser, éduquer à un usage mesuré et responsable du numérique. Éduquer est le meilleur investissement que nous puissions faire pour préserver notre planète. C'est la raison pour laquelle il faut intégrer dans la formation des enseignants un enseignement obligatoire à l'utilisation responsable des outils numériques. Je profite de cette prise de parole pour saluer également le travail du Sénat- celui de mon collègue Jean-Michel Houllegatte, mais également du président Patrick Chaize et du corapporteur Guillaume Chevrollier -, qui démontre que notre chambre

Alors qu'environ 80 % de l'empreinte environnementale du numérique provient des terminaux, la limitation de leur renouvellement constitue une question centrale pour maîtriser cet impact. Sans entrer dans les détails techniques de leur fabrication, il nous semble utile que les élèves prennent conscience de l'impact environnemental des biens numériques qu'ils utilisent. Le présent amendement tend à supprimer la mention relative aux usages, afin d'élargir la formation prévue à cette thématique et d'inciter les élèves à limiter le renouvellement de leurs terminaux et à adopter des comportements responsables dans leurs achats et de bonnes pratiques, telles que l'entretien et la réparation des appareils ou encore le recours au réemploi. Quel

doit porter sur l'impact environnemental des usages du numérique, afin de ne pas focaliser le contenu pédagogique sur la seule utilisation, c'est-à-dire ce que l'on fait avec l'appareil lorsqu'il est allumé. La notion d'usage permet, au contraire, de viser la façon dont on utilise physiquement l'appareil. Cette notion plus large englobe ainsi la mise en veille des équipements la nuit, le choix d'un matériel réparable ou reconditionné, le fait de limiter le renouvellement

Éric Gold. Prévue à l'article 2, la généralisation des modules relatifs à l'écoconception de services numériques au sein de la formation des ingénieurs en informatique est pertinente. Plus des trois quarts de l'empreinte environnementale du numérique provenant des terminaux, il convient également d'insister sur la formation des ingénieurs en matière d'écoconception des biens comportant des éléments numériques. Quel est l'avis de la commission

l'écoconception aux fournisseurs de données les plus importants, mais qui tend aussi à créer un référentiel. Il faut que ce référentiel, qui traduit une volonté politique,

des sites internet, des outils de communication électronique, est importante. C'est, en quelque sorte, prendre le sujet à la racine que

le Gouvernement est réservé, car il nous semble que la disposition est, à la fois, trop ciblée pour être introduite dans la loi et assez largement assez largement satisfaite par une mesure qui vient d'être adoptée dans la loi de programmation de la recherche, promulguée le 24 décembre dernier. Je parle de l'article 41 de cette loi, qui a permis d'inscrire dans le code de l'éducation la sensibilisation et la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable. A ainsi été inséré un 4° après le 4 de l'article L. 123-2 du code de l'éducation : le service public de l'enseignement supérieur contribue « à la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable

mais aussi d'étudier les gains apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire. Afin de prévenir les influences et les biais, le présent amendement prévoit que le décret d'application de cet article précise les modalités de composition et de fonctionnement de l'observatoire de manière à garantir son indépendance et son impartialité. Par ailleurs, il précise que la composition de l'observatoire doit comporter obligatoirement des membres choisis en raison de leur expertise en matière d'études d'impacts environnementaux du numérique et de transition écologique et solidaire. Ces conditions nous semblent nécessaires pour garantir la qualité de l'expertise.

est indépendant et que les personnalités qualifiées et les chercheurs qui le composent sont nommés en raison de leur expertise en matière d'impact environnemental du numérique et de transition écologique et solidaire ne semble pas concrètement

indique clairement que ses propres travaux ne peuvent se substituer à une évaluation complète de l'ensemble des impacts, qu'ils soient environnementaux, sanitaires, économiques, financiers ou sociaux.

proposition de loi. Je rappelle que l'article 24 permet de conditionner l'attribution des licences pour les nouvelles fréquences à l'impact environnemental. Concernant le cas spécifique de la 5G, une

sur les usages numériques et sa capacité à réduire l'impact environnemental. Je prendrai un exemple. Je me suis rendu cette semaine avec le président Richard Ferrand en Bretagne, nous avons visité une exploitation agricole qui avait poussé assez loin la numérisation de ses outils et de son fonctionnement. Grâce aux outils numériques, elle a par exemple diminué de 10

dans les « plus » et dans les « moins ». Pour reprendre la déclaration de M. le secrétaire d'État, il est tout à fait pertinent d'évaluer un impact non pas d'une manière subjective, uniquement dans les « moins », mais également dans les « plus » : d'où cette proposition qui paraît tout à fait justifiée.

par lettres en date des mardis 5 et 12 janvier 2020, le Gouvernement demande l'inscription le mercredi 27 janvier, après-midi et le soir, après les questions d'actualité au Gouvernement, sous réserve de son dépôt et de sa transmission, du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. En conséquence, l'examen des projets de loi autorisant la ratification du protocole à la convention relative relative aux infractions survenant à bord des aéronefs et autorisant l'approbation de l'accord entre la France et les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, est reporté au jeudi 28 janvier matin, en premier point de l'ordre du jour. Le Gouvernement demande également l'inscription, le jeudi 4 février, matin, en premier point de l'ordre du jour, du projet de loi autorisant l'approbation de la décision du Conseil du 14 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et l'après-midi, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ou de sa nouvelle lecture. Acte est donné de ces demandes. En ce qui concerne le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le délai limite de dépôt des amendements de séance pourrait être fixé le mercredi 27 janvier à pour la première lecture, et le jeudi 4 février à l'ouverture de la discussion générale en cas de nouvelle lecture. En cas de nouvelle lecture, la durée de la discussion générale pourrait être fixée à quarante-cinq minutes. Y a-t-il des observations ?